la séance est reprise, nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2023. Et dans la suite de la discussion de la mission Santé : la parole est à Madame Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains, madame la présidente. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues, à quoi sert la mission Santé certainement pas a donné le cap et à financer la politique publique du même nom, d'abord parce que dans notre pays, la santé est très largement financé par l'assurance maladie, ensuite parce que les orientations sont donnés par le ministère de la Santé, dont les directions financé par le programme, support de la mission Solidarité que nous venons d'examiner ces orientations, enfin, sont exécutés par le système des agences sanitaires qui, au fil des débudgétisation ne sont plus financées que de façon résiduelle par la mission Santé, seul l'Institut national du cancer, l'Office national des accidents médicaux ou Ankara encore la part du financement de lancer ce qui revient au ministère de la santé ont résisté à ce mouvement de transfert vers l'assurance maladie. La Haute autorité de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament ou encore l'Agence nationale de santé publique sont désormais financés à 100 % par la Sécurité sociale, le bilan de ce qui était au départ une simplification par le décroisement des dotations et une garantie pour les gestionnaires par l'assurance que leurs dotations échapperait à la régulation budgétaire hé bien négatif pour les parlementaires et les citoyens, c'est l'opacité de la boîte noire de l'Ondam objectif national d'assurance-maladie, quand ce n'est pas comme pour Santé publique France un détournement complet du principe de l'autoradio l'autorisation budgétaire qui permet de dépenser plusieurs milliards d'euros sans en rendre compte, tout en en faisant partiellement retour au budget de l'État, on comprend que cette souplesse soit apprécié, mais elle ne nous semble pas admissible de surcroît le changement de financeurs n'est pas neutre pour les agences gestionnaire me faisait récemment part de sa difficulté à négocier ses effectifs avec Bercy et le reste avec la CNAM, sans que le résultat final ne tiennent forcément compte des différents engagements pris la programmation des stocks d'équipements de protection des vaccins n'est pas l'affaire de l'assurance maladie et c'est normal, la mission santé est donc devenue la mission de l'aide médicale d'État, il est tout à fait légitime de s'intéresser à ce dispositif, qui mobilise des moyens considérables, mais il ne saurait constituer à lui seul une politique de santé, ce ne sont pas les quelques actions de prévention sanitaire qui viennent infirmer ce constat une nouveauté cette année, la mission Santé fait transiter des fonds européens vers le volet investissement Ségur du plan de relance français je ne suis pas certaine que cette voie de cette fonction de boîte aux lettres suffisent à justifier l'existence de la mission à défaut d'une rebudgétisation du financement des agences sanitaires que nous privilégions en application du principe qui paie décide occupait pilote, il nous semble que l'existence de la mission Santé n'est plus justifié et que l'aide médicale d'État pourrait tout aussi bien trouver sa place au sein de la mission Solidarité alors que vous réfléchissez à la réforme de votre ministère, madame la ministre, je vous demande de considérer sérieusement cette question loin d'être anodine pour qui veut construire, conduire une politique de santé dans notre pays sous le bénéfice de ces observations, le groupe les Républicains se prononcera néanmoins en faveur des crédits d'émission sous réserve de l'adoption des amendements proposés par la commission des finances et la commission des affaires sociales, je vous remercie. Merci madame la présidente, la parole est à Madame Véronique Guillotin, pour le groupe RDSE.

l'examen de la mission santé du PLF et depuis quelques années, l'occasion de constater le caractère chétif éparses des crédits qui lui sont consacrés, en effet, s'agissant des dépenses de santé qui ne figure pas dans le PLFSS nous sommes face à un budget au périmètre limité : 3 4 milliards en autorisations d'engagement et en crédits de paiement contres les 600 milliards de la Sécurité sociale, cette année, pourtant un nouveau programme, voit le jour au sein de cette mission que nous disions tout son déclin, ce programme 379 consacré au soutien européen, l'investissement dans les établissements de santé et aux dons de vaccins aux pays étranger devient ainsi le plus cher de la mission avec un budget de près de 2 milliards d'euros, il doit notamment permettre jusqu'en 2000 26 de recueillir et transférer les 6 milliards de crédits européens sur le volet investissement du Ségur de la santé destiné aux établissements de santé aux établissements médico-sociaux et à l'amélioration des outils numériques en santé 800 établissements vont être soutenus dans leurs investissements du quotidien, ainsi que 20 projets de construction modernisation ou rénovation énergétique dont le montant est supérieur à 20 millions d'euros quand on connaît le niveau de dégradation de nos établissements qui participent à la dégradation de l'accueil des patients, mais aussi des conditions de travail de nos soignants, ces sommes sont particulièrement les bienvenues, leur présence dans la mission santé du PLF nous permettra par ailleurs de contrôler la bonne utilisation de ces crédits opération plus délicate s'il se perdait dans le budget colossal de la sécurité sociale, le 2ème poste de dépense, le plus important de la mission, et celui de l'aide médicale d'État, évaluée à 1,14 milliards d'euros en 2023, en hausse de 10 rappelons que le gouvernement depuis le quinquennat précédent, fait un effort de sincérité louable sur ces crédits, les modifications législatives et réglementaires de 2019 visant à limiter les détournements du dispositif sont nécessaires mais reste difficile à évaluer, tant elles ont subi d'aménagement du fait de la crise Covid le retour à la normale, ou du moins l'abaissement du niveau de crise nous permettra peut-être d'en tirer des conclusions, l'an prochain, l'évaluation de nos politiques publiques et, bien sûr, une nécessité qui doit nous faire progresser vers un dispositif équilibré, le débat ne peut toutefois être déconnectée du contexte international, fait de crise de conflit de dérèglement climatique et donc de déplacements de population, l'épidémie mondiale que nous avons connu, nous rappelle aussi l'importance de prendre en compte ces dépenses comme partie intégrante de notre politique de santé publique, sous peine de voir émerger ou resurgir de très nombreuses, de très nombreux virus se contenter de la prise en charge de situation d'urgence un effet pervers, en effet, mieux vaut soigner une bronchite qu'une décompensation respiratoire et puis ce que l'on parle d'argent, cela coûte moins cher, méfions-nous des solutions faciles, d'autant qu'aucun médecin ne laissera sur le bord du chemin une personne qui en a besoin, comme personne d'ailleurs dans cet hémicycle, notre groupe ne votera pas l'amendement du rapporteur spécial, mais il sera favorable à l'amendement porté par Madame la rapporteure, s'agissant du programme 200 IV quelques actions en augmentation sont à noter sur le volet prévention celle consacrée à la nutrition santé environnementale, prévention des addictions ou encore le sport santé je veux redire ici que la nomination d'un ministre de la Santé et de la prévention est un signal positif qui doit être accompagné d'une véritable révolution de la prévention pour de nombreuses maladies si les facteurs de risque sont multiples : beaucoup sont aussi liés à leur mode de vie, nos habitudes alimentaires et bien sûr l'environnement c'est le concept de santé unique et je profite donc de cette tribune, Madame la Ministre, pour redire que les attentes sont fortes pour des investissements à la hauteur des enjeux et au plus près des besoins de chaque territoire s'agissant du vote de la mission, notre groupe se déterminera en fonction du sort réservé aux différents amendements. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Agnès Firmin Le Bodo Ministre délégué chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé, Madame la Ministre. Madame la présidente, madame la rapporteure pour avis, monsieur le rapporteur spécial, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les sénateurs, je me réjouis de présenter devant vous, l'émission, les crédits de la mission santé en parallèle du budget de la Sécurité sociale, l'examen de cette mission constitue toujours un moment important du calendrier parlementaire, davantage peut-être que d'autres missions du budget de l'État, la mission Santé reflète nos interrogations collectives et la nécessaire réponse de la puissance publique pour prévenir et anticiper les besoins en santé de nos concitoyens, la pandémie a constitué en ce sens un révélateur, elle nous a douloureusement rappelé les Liens entre santé humaine santé animale et biodiversité : les crédits de la mission santé en complément du budget de la Sécurité sociale concrétise les priorités du gouvernement pour mieux protéger nos concitoyens et faire face à ces défis nouveaux la santé environnementale constitue une priorité de ce gouvernement, mieux comprendre et tenir compte des Liens entre santé humaine et notre environnement est aujourd'hui essentiel, cela se traduit par la poursuite et l'approfondissement des différents plans déjà engagés comme le Plan national santé environnement IV, le gouvernement entend également porter une politique ambitieuse pour la santé des femmes, je pense à la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose ou l'extension du remboursement de la pilule du lendemain pour toutes les femmes, l'ambition du gouvernement c'est ainsi celle d'une véritable politique en matière de prévention à travers plusieurs mesures. D'abord avec de nouveaux rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie prévue en Plfss pour 2023, c'est un enjeu décisif pour lutter contre les inégalités en santé, il s'agit ensuite de l'élargissement du dépistage sans ordonnance et de sa prise en charge à 100 % pour les moins de 26 ans à d'autres IST que le VIH l'extension à d'autres professionnels de santé, des possibilités de prescription des vaccins recommandés par le calendrier vaccinal, enfin, c'est un effort renouvelé en matière de prévention avec l'augmentation du prix du tabac pour lutter contre le tabagisme, première cause de mortalité évitable et de mortalité par cancer en France, en complément de cette dynamique, ambitieuse dans le budget de la Sécurité sociale, les crédits du programme 204 participe de l'action de l'État pour mieux anticiper et protéger nos concitoyens. Il vise à améliorer l'état de santé général de la population dans un souci de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé avec la mise en place de plans et de programmes de santé pilotée au niveau national, la sécurité sanitaire est également un Champ important du programme, afin de garantir la protection de la population face à des événements sanitaires graves menaçant la santé de la population, comme en témoigne la pandémie de Covid 19 19 3 objectifs figurent dans ce programme, prévenir le développement de pathologies le plus en amont possible, comme par exemple avec la campagne de vaccination contre la grippe, qui est aujourd'hui engagée, elle démarre d'ailleurs assez timidement donc vaccinez-vous et encouragé à se faire vacciner, assurer à toute la population, un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire comme, par exemple, avec le soutien de l'Agence Régionale de Santé à Wallis et Futuna, préparer, coordonner et piloter les opérations de gestion et de Cristiani terre en lien avec l'ensemble des institutions et opérateurs impliqués et en anticipation stratégique des risques comme par exemple le financement du système d'information comme le le logiciel et si qui concourt à la mise en oeuvre, le suivi et le pilotage de la campagne vaccinale contre la Covid 19. La mission Santé reflète également l'engagement de fraternité envers les plus démunis qui est au coeur de la promesse républicaine: l'aide médicale d'État répond à cette exigence forte de solidarité et de générosité, le programme 183 protection maladie assure en effet en en complément des politiques de sécurité sociale, la protection face à la maladie dans des situations relevant de la solidarité nationale, il vise essentiellement à financer l'aide médicale d'État AME dont la gestion est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie avec un double objectif humanitaire et sanitaire en direction des publics les plus défavorisés, instaurée en 2000 l'AME de droit commun, hein, sur un si la protection de la santé des personnes étrangères de démunis vivant en France en situation irrégulière vis-à-vis du droit au séjour et ne pouvant donc être pris en charge par la protection universelle maladie, elle protège les personnes concernées en leur permettant l'accès aux soins préventifs et curatifs et joue un rôle important en matière de santé publique, en évitant que les affections contagieuses non soignées ne se propage, enfin, elle permet de faciliter la prise en charge des soins en amont, évitant ainsi pour nos établissements de santé des gens en souffrance, les surcoûts liés à des soins retardés et pratiqués dans l'urgence, depuis 2020, le gouvernement a mis en place des mesures pour d'une part, accentuer les efforts sur la gestion du positif et la régulation de leurs dépenses et, d'autre part, renforcer les contrôles dans le cadre de programmes d'action ambitieux. En 1er lieu les programmes de centralisation de l'instruction des demandes d'AME et de traitement des factures de soins urgents ont renforcé l'efficience du dispositif en dégageant des gains financiers grâce à une gestion plus efficace, en second lieu, afin de veiller à la juste attribution de l'AME et de garantir l'accès aux seuls ayant droit, la lutte contre les abus et les détournements Xisco positif a été renforcée pour cela plusieurs j'actions ont été engagées, l'obligation de déposer une prime demande d'AME en personne à la CPAM la détection des dissimulations de visas grâce à l'outil visa bio qui permet de vérifier si les demandeurs ne dispose pas de VISA, auquel cas il serait en situation régulière et donc nous, on est Gilles l'application d'un délai d'ancienneté à l'AME de 9 mois pour la délivrance de certaines prestations programmées, la demande d'un accord préalable du service du contrôle médical de la CPAM pour les cas les plus urgents. L'année 2023 sera consacré au suivi de ces mesures de renforcement des contrôles qui n'ont pu être mis pleinement en oeuvre durant la crise Covid aucune majorité n'a remis en cause l'AME depuis sa création, parce qu'elle constitue en réalité une mesure de bonne gestion des deniers publics et un outil sanitaire essentiel, le gouvernement se posera ainsi fermement à toute initiative visant à remettre en cause le périmètre des soins couvert par l'AME sans naïveté ni angélisme dans la lutte contre les éventuels abus mieux répondre aux besoins aujourd'hui de notre système de santé tout en anticipant les défis à venir cet enjeu s'inscrit dans la démarche du Conseil national de la refondation en santé qui est décliné actuellement dans les territoires, c'est bien à partir du terrain et des initiatives des acteurs avec l'accompagnement de l'État que nous construirons la santé de demain en renforçant l'accès aux soins dans une logique de confiance, de coopération et de subsidiarité, je vous remercie. Merci madame la ministre. Je vous rappelle que pour cette mission, la conférence des présidents a fixé la durée maximale de la discussion à 2 en conséquence. Si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à 23 heures 20, celui-ci se poursuivrait à la fin d'émission de cette semaine et nous passerions à l'examen de la mission, plan de relance, je vous rappelle que nous avons 32 amendements à examiner, en revanche, si nous terminions avant le terme de cette durée, l'examen de la mission suivante pourrait commencer sans attendre, nous allons donc procédé à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Santé figurant à l'état B. par nous commençons, pardon, par 15 amendement faisant l'objet d'une discussion commune, à commencer par l'amendement présenté par Monsieur Klinger, au nom de la commission des finances 24. Merci madame la présidente, la commission des finances propose une réduction de 350 millions d'euros des crédits proposés pour la émeut pour plusieurs raisons, que j'ai évoquées dans mon intervention liminaire premièrement, le gouvernement justifie le montant des crédits par la prolongation de l'évolution tendancielle, observée avant la crise sanitaire, c'est-à-dire une progression continue du nombre d'étrangers en situation irrégulière, cela nous paraît très problématique, quelques semaines avant le dépôt d'un projet de loi censée maîtriser les flux migratoires et faciliter la reconduite aux frontières, deuxièmement, nous constatons que les mesures de contrôle et de lutte contre la fraude, qui avait été présenté il y a 3 ans, en réponse au constat dressé dans les rapports des inspections des affaires sociales et des finances ont été peu efficace, elle mériterait d'être renforcée 3ème point le niveau des crédits demandés est supérieur de près de 200 millions à celui des dépenses de 2022 établie dans le PLFR voté la semaine dernière, ce serait une augmentation de 20 % d'une année sur l'autre peu justifiable d'autant que l'État est en situation de créanciers vis-à-vis de l'assurance maladie, ce qui est nouveau par rapport aux années antérieures, enfin, la commission propose au Sénat de reprendre l'amendement qu'il avait adoptée il y a 2 ans pour redéfinir la émeut et aligner son périmètre sur celui constaté dans la plupart des autres pays européens voisins cette évolution de l'AME comme des mesures de contrôle plus effective et une meilleure maîtrise de l'immigration irrégulière, permettrait de ramener les dépenses d'AME en dessous de 900 millions d'euros, comme le propose notre amendement. Merci, monsieur le rapporteur, nous passons 665 rectifié madame mon. Merci madame la présidente par cet amendement, nous demandons au gouvernement, le lancement d'un plan d'urgence pour la psychiatrie depuis les années 1980 malgré une augmentation de la population générale, les moyens pour la psychiatrie ont non seulement peu évoluer mais ont souvent souffert de la fermeture de 2 tiers des lits d'hospitalisation, la psychiatrie, parent pauvre de la médecine est un secteur de plus en plus sinistré qui appelle à une refonte radicale que les A6 organisée par le gouvernement, n'ont guère pour une pour une prise en soins de qualité, il s'agit de renforcer les moyens pour permettre l'accueil des patients selon les besoins et les attentes d'améliorer les conditions de travail des soignants de lutter contres les mesures privatives de liberté, faute de moyens humains suffisants et de garantir en cela le respect des droits fondamentaux des des patients. D'investissement public dans la psychiatrie dont la pédopsychiatrie, proche de l'effondrement, doit permettre l'ouverture de lits nouveaux et de structure ouverte pour accompagner les patients et permettent le recrutement et la formation de personnel qualifié cet amendement crée donc un nouveau programme intitulé Plan d'urgence pour la psychiatrie, doté de 1 milliard d'euros aujourd'hui pour la 2ème fois cette année, 4 syndicats appelaient à une journée de mobilisation et de grève, il est temps, Madame la Ministre, de les entendre. Merci madame la présidente, alors par cet amendement, nous proposons d'allouer des crédits pour la compensation de l'inflation, notamment énergétiques et alimentaires pour les accueils de jour autonomes, l'accueil de jour, propose un accompagnement personnalisé aux personnes accueillies et un soutien aux aidants, et aux attentes selon l'Insee, en septembre 2 22, les prix à la consommation ont augmenté de 5 6 pour 105 6 % sur une durée d'une année d'ailleurs un peu plus en octobre dans le médico-social, la situation et tout autant difficile et l'inflation pèse sur les structures qui déjà se trouvent en manque de financement pour simplement parvenir à l'équilibre, c'est pourquoi cet amendement propose de compenser les coûts de l'inflation pour les accueils de jour autonomes offrent domiciliaire par excellence, les accueils de jour autonomes représentent 24 % des places d'accueil de jour, les Epad donc 76 % les places d'accueil de jour représente donc autonome 32 de leur équivalent Epad et la somme qui a été consenti aux Epad comme bouclier énergétique relatifs au gaz étant de 1 milliard d'euros pour le 2ème semestre 22 par une simple règle de 3, cet amendement vise à compenser l'inflation pour les accueils de jour, de 1000 autonome à hauteur de 320 millions d'euros, donc nous avons dû bien sûr diminuer les crédits de l'action en plus aide médicale d'État, et donc de ce fait, nous nous, ça peut long à lever le gage. Merci, cher collègue, le 522 rectifié Monsieur dessus. Merci madame la présidente, aujourd'hui, l'accès à l'aide médicale d'État est réservée aux personnes résidant depuis plus de 3 mois en France et ne disposeront pas de titre de séjour, les raisons de ce délai, instaurée par le décret du 30 décembre 2019 sont à la fois budgétaire mais aussi et surtout il budgétaire pour faire des économies sur la misère, c'est une constante de ce gouvernement et on vient de le voir de la majorité sénatoriale également mais surtout idéologique pour ne pas employer un autre mot car étrangement pour les réfugiés ukrainiens, ce délai n'a plus lieu d'être, et ils ont accès à la couverture santé dès leur entrée sur le territoire, ce qui est louable mais le double jeu et tout de même assez scandaleux au delà de l'aspect éthique de l'aide trois mois est un non-sens économique et sanitaire, économique, car en créant des obstacles à l'accès aux soins et à la santé d'un public déjà fragilisé, on n'efface pas la maladie, un non-sens sanitaires collectifs puisqu'au-delà de la solidarité, c'est toute la population française ou la santé peut être fragiliser si les maladies venus d'autres pays ne sont pas traitées à temps et se propage par la suite, voilà pourquoi nous proposons une hausse du montant accordé à l'AME de 10 %. Merci le 664 Madame Poncet, monde. Merci madame un président à heure les établissements de santé médicaux sociaux représentent annuellement 2 % de la consommation énergétique nationale, plus de 700000 tonnes de déchets 1,5 milliards de repas 401200 litres d'eau par lit et par jour, le rapport du groupe de réflexion The Shift Project, estime la contribution du secteur de la santé aux émissions de gaz à effet de serre à 8 % du total national la vétusté d'une partie du Patrimoine et les consommations d'énergie particulièrement important des établissements les rendent ainsi vulnérable aux difficultés d'approvisionnement en énergie et hausses massives de tarifs annoncées, il est donc nécessaire de donner les moyens aux établissements de santé et médico-sociaux de relever le défi de la transition énergétique et écologique, le fonds pour la transition écologique du système de santé est ainsi destiné à accompagner les projets de transformation énergétique écologique des établissements sanitaires et médico-sociaux, l'amendement, abonde un nouveau programme font pour la transition énergétique et écologique du système de sentiers de santé de 50 millions d'euros.

prévoit la création d'un nouveau programme dans la mission Santé intitulé carte Vitale biométrique et doté de 20 millions d'euros, l'amendement adopté en juillet dernier, je dis bien juillet dernier au Sénat sur l'initiative de notre groupe avait reçu un avis de sagesse du gouvernement qui avait même levé le gage, il avait été retenu dans le texte définitif à la suite de l'accord obtenu en commission mixte paritaire avec les députés, ce nouveau programme devait être le numéro 378 vous voyez, il est précis, figurer dans le projet de loi de finances pour 2023, pourtant il n'en est rien, le programme 3 78 a disparu du bleu budgétaire et aucun crédit n'est prévue pour lancer le chantier de la carte Vitale biométrique le lancement du chantier ne souhaite de nouveau repoussée dans l'attente d'expérimentation qui ne cesse de succéder sans aucune prise de décision, mais au-delà du fond et de, je ne le j'ai évité d'ailleurs de relancer le débat sur la pertinence de la carte biométrique, Madame la Ministre, mon intervention concerne surtout la méthode du gouvernement qui consiste à prendre une position au mois de juillet, et quelques mois plus tard, de changer diamétralement de position avec une vision sans explication, sans groupe de travail sans mission au regard des engagements qui ont été pris, Madame le Ministre, cette méthode de relations avec le Sénat est particulière et en tous les cas, votre prise de position aujourd'hui, nous, on nous montrera quelle façon de travailler, vous voulez demain matin avec le Sénat, merci. Merci, chers collègues, nous passons trois. 328 présenté par Madame la rapporteure au nom de la commission des affaires sociales. Merci madame la présidente, madame le Ministre dans un souci de maximisation de l'accès aux soins et à la prévention des bénéficiaires de l'aide médicale de santé publique, le présent amendement crée au sein de la mission Santé un programme consacré au financement d'actions conduites par l'État, l'assurance maladie et les associations, notamment dans le cadre de démarche d'aller vers telle que les maraudes des bus de prévention ou encore des barnums de dépistage afin de proposer des examens aux personnes en situation irrégulière et de les sensibiliser sur la nécessité de solliciter le dispositif de l'aide médicale de santé publique pour bénéficier d'examens complémentaires de prévention, il est prévu de transférer 10 millions d'euros du programme 183 vers ce nouveau programme, ce transfert ne devrait pas avoir d'impact sur la soutenabilité des dépenses du programme 183 compte tenu des économies appelé à découler du renforcement des contrôles et du recentrage du panier de soins de la nouvelle aide médicale de santé publique. Merci madame la rapporteure, nous passons 677 il est présenté par Madame Jasmin. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer un nouveau programme dédié à la santé mentale et à le doter de 10 millions d'euros pour l'année 2023 les troupes psychique concerne chaque année un Français sur 5 et leur prise en charge constitue le 1er poste de dépenses de l'assurance maladie depuis là devant la prise en charge des cancers cet enjeu de santé publique majeur a pris une forte résonance pendant la crise, la crise depuis maintenant 3 ans, nous subissons évidemment les effets le climat anxiogène d'des certitudes et des mesures de restriction qui ont accompagné cette crise cette crise affecte la santé mentale de grand nombre de nos concitoyens dans la vie sociale et parfois la situation économique se sont troublés par ailleurs bouleversé, se sont trouvés ma par ailleurs certains publics, notamment les jeunes sont particulièrement touchés, et c'est dans ce contexte que mon collègue Jean Sol et moi-même avons fait au nom de la commission des affaires sociales, rapport d'information numéro 3 sur les effets de l'épidémie sur la santé mentale, ce nouveau programme et donc la traduction de la priorité collective que nous souhaitons donner à notre système de santé mentale pour mieux prendre en charge nos concitoyens merci. j'ai eu l'occasion de leur présenter une autre mission, il a été retoqué, donc il est inscrit cette mission santé la médecine intégrative et quelque chose de particulièrement intéressant, en plus de la médecine traditionnelle, elle permet de prendre en compte : le patient dans toute sa dimension à la fois social professionnel et le but de cet amendement, c'est de prendre la le côté préventif notamment ou prescriptif en tout cas de la médecine intégrative, pour faire en sorte qu'il y ait des programmes de recherche qui permettent qu'elle se développe comme elle se développe dans des pays étrangers, c'est la raison pour laquelle nous proposons une somme de 5 millions d'euros, qui est pris sur un autre programme pour faire en sorte de développer en France, la médecine intégrative. Merci, cher collègue, nous passons à l'amendement 620 Madame Poncet mange. Merci madame la présidente, alors cet amendement que le groupe écologiste propose porte propose d'améliorer le Nutriscore on incluant l'impact environ environnementale dans ses critères de notation le Nutri score est un 1er pas dans la bonne direction pour encourager à mieux manger, mais il a ses limites, d'abord, il n'est pas présent sur tous les les produits il est facultatif, ensuite il ne prend pas en compte l'impact environnemental de chaque produit dans le rapport de mars 2022, issu de la mission d'information, protéger protéger et accompagner les individus en construisant la sécurité sociale, écologique du XXIe siècle que Mélanie Vogel a eu le l'honneur de porter, nous avons proposé cette amélioration, il faudrait d'abord opéré une distinction entre produits bruts ou peu transformés et aliments ultratransformés ceci ont un impact plus délétères sur la santé mais également sur l'environnement, une banane n'a pas le même impact sur votre santé qu'un gâteau à la banane, bourré d'addictif, mais elle peut avoir un impact sur l'environnement, si elle est ramenée depuis l'autre bout du monde hors saison, de sa culture, or la dégradation du climat et de la biodiversité est en lien Direct avec notre capacité collective à mieux nous nourrir, si nous n'avons plus de sol fertile, si nous avons des sécheresses terrible tous les étés des inondations tous les automnes notre capacité à nous nourrir sera gravement dégradée, nous proposons donc cette amélioration du nutriscore afin que chacun puisse choisir des produits bien notée tous notés en sachant ce qui est bon pour soi mais aussi pour la planète. Merci, nous passons 129 rectifié bis et Madame Imbert qu'présente merci. Si madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, malgré des avancées considérables, le virus du SIDA et les infections sexuellement transmissibles en général demeure de véritables drames et une vraie préoccupation en matière de santé publique aussi les fondamental de poursuivre la lutte contre ces maladies, cet amendement est inspirée par le rapport que j'avais remis au nom de la commission des affaires sociales du Sénat, en juillet 2019 à la suite d'une enquête de la de la Cour des comptes et ce rapport s'engager pour un avenir sans SIDA met en lumière une épidémie cachée mentionnant : plus de 30000 personnes malades non prise en charge et responsable de plus de 60 % des nouvelles contaminations dans le cent

juste pour dire que, parmi les recommandations de de ce rapport, hein s'engager pour un avenir sans SIDA, il est proposé d'encourager la recherche pour des schémas thérapeutiques aisément observables, donc, cet amendement vise à augmenter les crédits en faveur de la prévention du VIH et des IST à hauteur de 3 millions d'euros Crédit prélevés sur l'action de aide médicale de l'état du programme 183 pour abonder l'action 14, prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades du programme 204 et donc je reviens si vous le permettez à l'amendement suivant.

latérale latérale amyotrophique, plus connu sous le nom de maladie de Charcot demeure un drame et nous le savons tous pour les personnes touchées et pour leurs familles, qu'on en parle de plus en plus cette pathologie est encore trop méconnue, dans le domaine de la recherche et les traitements actuels demeurent trop insuffisant cet amendement on voit plus qu'un signe pour que la sclérose latérale amyotrophique devienne elle aussi une cause nationale, parmi les 7000 maladies rares recensés la maladie Charcot est une des maladies la la plus fréquente cette maladie neuro-dégénérative terrible, incurable, doit nous mobiliser et nous devons renforcer la recherche sur cette maladie, donc, cet amendement vise également augmenter les crédits en faveur de la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, à hauteur de 3 millions d'euros. Merci, cher collègue, nous passons 254 rectifié bis Monsieur Savary. Merci madame la présidente, alors là c'est un amendement qui concerne la cryothérapie corps entier, il y a une différence, c'est pas la cryothérapie qui risque de griller les tégument hein la la cryothérapie corps entier qui est encore très méconnue dans notre pays et qui permet d'améliorer les troupes du sommeil, de réduire la douleur ou encore de réduire l'anxiété, elle est également un allié dans le processus d'année, amélioration de la fonction respiratoire, nous avons été sensibilisés avec Corinne Imbert parce qu'il y a des jeunes qui sont investis là-dedans et véritablement c'est un progrès tout à fait significatif et, au-delà de sa prise en charge orienté sur l'accompagnement de différents besoins récupération sportive, amélioration du bien-être, l'amélioration de la qualité de la vie, l'accueil Rio thérapie corps entier se développe à travers des pôles de recherche des comités scientifiques qui sont composés de différents acteurs de santé dont de grands professeurs de médecine, par expérience, expertise des travaux de recherches actuelles ainsi que les protocoles de prise en charge, souligne l'absence d'effets secondaires négatifs et met en avant l'absence d'atteinte aux tégument lors d'une séance de cryothérapie corps entier en immersion complète, il faut faire encore là-dessus des recherches tout à fait indispensable, c'est la raison pour laquelle nous proposons une somme de 500000 euros sur le compte prévention merci.

qui ne peut être présent aujourd'hui, c'est un sujet qui lui est cher et qui a fait l'objet d'une plus âgé, en octobre dernier sur le territoire des îles Wallis et Futuna, le système de santé local repose sur une agence de santé créer par ordonnance en 2000 et qui est chargé de l'élaboration du programme de santé du territoire, de sa mise en oeuvre et de la délivrance des médicaments, c'est un établissement public national administratif disposant de l'autonomie administrative et financière et là, sur la protection sanitaire du territoire et de ses 120000 habitants, elle perçoit notamment une dotation versée par l'État au sein du programme de 204 de la mission Santé ce rappel institutionnel nous emmène au sujet de cet amendement. L'insuffisance rénale à Wallis le et Futuna, il est, elle est prise en charge par cette agence, via une convention avec une association néo-calédonienne, le centre de dialyse possède une capacité d'accueil maximale de 35 patients alors que qu'une centaine de personnes attendent aujourd'hui de se faire soigner après plus de 10 ans d'attente, un centre d'hémodialyse est en cours de construction à Futuna mais il ne sortira pas de terre dans les délais prévus, de plus, il ne sera doté que de 4 postes pour répondre aux besoins d'une population qui aujourd'hui doit s'exiler à Nouméa pour se soigner, chers collègues, les dialysés de Wallis et Futuna, sollicite l'accès à un traitement digne à des soins de qualité, en attendant que les besoins de la population dialysé qui a triplé en 10 ans, soit réellement prise en compte cet amendement propose de remplacer en urgence les 8 générateurs d'hémodialyse obsolète, ainsi que l'achat de véhicules pour le transport des malades, il vise aussi à augmenter les crédits à hauteur de 450000 euros pour les dialysés de Wallis et Futuna, poulet aux familles pour ce territoire français de l'autre bout de la terre, je vous demande chers collègues

Merci madame la présidente, cet amendement d'appel vise à renforcer considérable considérablement les moyens alloués à la prévention en santé mentale en France, les troubles anxio-dépressifs et cognitifs ont fortement augmenté avec la crise liée à la pandémie de Covid 19 ils ont notamment affecté la jeunesse et risque de marquer durablement l'avenir de nos sociétés, les coûts sociaux économiques de ces pathologies sont considérables, une espérance de vie réduite de 15 à 20 ans en France la sentimentale et le 1er poste de dépenses de l'assurance maladie, avec 19 milliards trois d'euros par an devant les cancers et les maladies cardio- vasculaires, pourtant la santé mentale demeure le parent pauvre de notre système de santé, le financement de la recherche publique en psychiatrie ne représente que 2 à 4 pour 100 du budget de la recherche biomédicale en France soit la des plus faibles des pays européens, même constat pour les carrières médicales, près de 30 % des postes de psychiatres sont vacants en France et les maladies mentales sont sans doute l'un des derniers tabous sociaux. La parole ne sait pas encore libéré à ce sujet, les besoins d'accompagnement mentale sont forts et nombreux nécessite donc des investissements massifs et des politiques publiques d'envergure et, notamment, des moyens supplémentaires pour prévenir l'apparition pour prévenir l'apparition des symptômes dépressifs, malheureusement les moyens prévus par la mission santé demeurent largement insuffisant pour répondre aux besoins de la population notre amendement proposant de financer un nouveau programme consacré à la prévention en santé mentale, doté de 200000 euros en 2023, telle est le sens de cet amendement d'appel. Si merci, cher collègue et nous passons à la vie de des de la commission, monsieur le rapporteur Merci madame la présidente, non pour l'amendement 665 un avis défavorable, la prise en charge des troubles psychiques et, bien entendu, un un enjeu majeur de santé publique et le secteur de la psychiatrie est actuellement en difficulté, les questions de financement soulevés sont toutefois du ressort de la sécurité sociale et non d'une ligne budgétaire psychiatrie sur la mission Santé au surplus l'amendement supprime la quasi-totalité des crédits de l'AME, ce qui ne paraît pas réaliste pour l'amendement 663 avis défavorable car le financement des structures d'accueil de jour et donc de leurs charges de fonctionnement ne relève pas de l'État, l'amendement 522 avis défavorable puisque la commission des finances souhaitent un recentrage de l'aide médicale d'État sur les prises en charge comparables à celles prévues dans la plupart des pays européens voisins pour les étrangers en situation irrégulière. Amendement 664 avis défavorable, le plan d'investissement pour les établissements de santé et des établissements médico-sociaux comportent une importante dimension énergétique et écologique, c'est d'ailleurs une condition pour bénéficier du soutien des fonds européens, qui représentent, je le rappelle 6 milliards sur 5 ans pour l'investissement en santé, la création d'un fonds spécifique ne paraît donc pas nécessaire. L'amendement 212, le Sénat a créé le programme carte Vitale biométrique dans la loi de finances rectificative d'ce dernier le gouvernement avait d'ailleurs levé le gage sur cet amendement, il est surprenant qu'aucune décision n'a été fournie sur les raisons de la disparition de ce programme dans le PLF pour 2023 née sur les actions engagées pour sécuriser l'usage de la carte vitale dans ces conditions, la commission des finances ne peut que maintenir la position adoptée l'été dernier. L'amendement 328 avis favorable, le Sénat avait adopté il y a 2 ans, un amendement identique de la commission des affaires sociales, il paraît en effet utile de pouvoir renforcer les actions de prévention en direction des personnes en situation de précarité, et plus spécifiquement l'espèce de celles d'entre elles qui sont en situation irrégulière, l'amendement 677 avis défavorable comme sur l'amendement 665 précédemment mentionnés, l'amendement 366 la définition de nouveaux types de prise en charge, tels que la médecine intégrative, me paraît relever avant tout des instances chargées d'évaluer les pratiques et d'établir des recommandations en matière d'organisation des soins et de prise en charge ce programme budgétaire ne me paraît pas être le vecteur le plus approprié, je demande le retrait de cet amendement donc retrait ou avis défavorable. Amendement 600 le Nutri score a été mis en place par Santé publique France avec l'expertise scientifique de ANC et du Haut Conseil de la santé publique, la France participe également aux travaux européens visant à étendre ce système d'étiquetage nutritionnel et à étudier ces évolutions possibles, il existe des débats scientifiques sur les modalités de calcul du score, c'est bien entendu un enjeu important sur lequel il faut continuer à travailler dans nos instances nationales comme au niveau européen, je ne suis pas certain que cela passe par la majoration de crédits qui est proposé : demande de retrait ou avis défavorable. Pour l'amendement 129 130 et 254 ces amendements soulèvent la question de la vocation du programme 200 et de la capacité de la direction générale de la santé à travers ce programme a réellement piloter des actions de prévention et de santé publique, beaucoup d'actions financées par ce programme sont extrêmement dispersé, pour des montants généralement faibles, si bien qu'elles paraissent loin de disposer d'une masse critique suffisante pour prétendre produire un réel impact sur la réalisation des objectifs de santé publique poursuivi. Une grande part des moyens financiers se trouve ailleurs, dans des organismes financés par l'assurance maladie, je souscris évidemment à l'objectif de ces un de ces amendements portant sur la maladie de Charcot, le VIH ou la cryothérapie corps entier, je suis en revanche plus réservé sur l'ajout de nouvelles actions dédiées à telle ou telle pathologie sur ce programme, alors que le pilotage de la recherche de la prévention lui échappe largement la commission des finances s'en est remis à la sagesse du Sénat sur ces trois amendements. L'amendement 700. La commission des finances souhaite connaître l'avis du gouvernement sur le problème très précis de l'hémodialyse à Wallis et Futuna, j'ajoute qu'une conférence territoriale de santé prévue prochainement, elle n'avait pas été réunis depuis 2005 et l'amendement 706 demandes de retrait ou avis défavorable sur cet amendement d'appel pour les raisons indiquées sur l'amendement proposant la création d'un programme psychiatrie. Merci, monsieur le rapporteur, madame la ministre, avis du gouvernement. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, tous ces amendements, on en point commun, ils portent un gage, maintenant je vais essayer sur des sujets aussi divers et variés, comme vous avez fait, monsieur le rapporteur, d'apporter l'avis du Gouvernement sur les amendements 24 et 522 tous les deux porte sur la il me l'souhaite augmenter les crédits, l'autre les diminuer, cela me fait penser que la proposition proposée par le gouvernement et la bonne qui allie à la fois l'enjeu d'humanité et l'enjeu de santé publique, donc un avis défavorable sur ces deux amendements l'amendement 663 qui porte sur l'accueil de jour, hein, demande de retrait ou un avis défavorable puisqu'il ne concerne pas du tout les crédits et l'objet dans le cadre de cette mission santé. Les amendements 665 et 677 et 706 un avis défavorable du Gouvernement concerne tous autour de la santé mentale, qui sont des enjeux nous partageons tous le point de vue que ce sont des enjeux importants, nous savons notamment que face à la crise sanitaire, les besoins de prise en charge en matière de santé mentale, mais aussi la nécessité de partager un état des lieux de la psychiatrie et de proposer des réponses aux difficultés identifiées, identifier les assises de la santé mentale et de la psychiatrie ont été organisées l'an dernier avec l'ensemble des acteurs. à l'issue de à l'issue de ces assises, le président de la République a annoncé un plan global pour la santé mentale, représentant au total un investissement de 1,9 milliards d'euros pour la période 2022 2026 2026 parmi les mesures phares de ces assises, en lien avec la promotion et la prévention santé mentale je retiens particulièrement les formation au secourisme en santé mentale qui ont fait leurs preuves pour améliorer les connaissances de tout un chacun sur les troubles psychiques les repérer ou reconnaître les signes précurseurs de crise afin d'éviter d'intervenir et d'éviter précocement ces formations déjà développé en milieu étudiant, pour être déployés dans tous les secteurs de la société et les 3 fonctions publiques devront être exemplaire à ce titre-comme le prévoit une circulaire interministérielle paru en février dernier, ce plan prévoit également l'accès facilité de tous un psychologue le renforcement déterminé de l'offre de psychiatrie hospitalière et ambulatoire des mesures fortes ciblée sur la pédopsychiatrie, mais aussi l'investissement dans la formation et la recherche en santé mentale le Ségur de la santé a également permis d'abonder financièrement le Champ de la psychiatrie publique notamment pour renforcer les CMP et les équipes mobiles de psychiatrie Pékin précarité, nous sommes donc déjà engagés dans la mise en oeuvre d'un plan d'ensemble pour revaloriser profondément la psychiatrie et je sais pouvoir compter sur la mobilisation des acteurs, notamment de la Commission nationale de la psychiatrie pour décliner cette politique nécessaire et ambitieux sur le territoire pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux amendements 559 665 677 et 706 l'amendement 212. Donc un avis défavorable du gouvernement, il concerne un gage. Pour développer la carte biométrique et abondé de 20 millions d'euros, des crédits de nouveau en 2023 alors que nous savons qu'une mission IGAS a été lancé que les crédits déjà votés en 2022 n'ont pas été voter et, donc, pouvoir continuer de pouvoir attends les résultats de cette mission IGAS et d'utile d'utiliser les crédits déjà votés en 2022 donc pas nécessaire de voter des crédits sur 2023 donc un avis défavorable, les amendements 366 et 254 qui concerne concernant la médecine intégrative et la cryothérapie, donc le fait de se mettre tout entier dans une bassine de glaçons, comme les font les sportifs et notamment les rugbyman. pas que mais aussi mais aussi donc la médecine intégrative hein est utilisé pour désigner le recours simultanée à la médecine dite conventionnelle, s'appuyant sur des traitements qui ont toujours obtenu une validation scientifique et aux médecines alternatives dans le suivi d'un patient, le gouvernement est particulièrement attentif au développement des pratiques de médecines alternatives ou non conventionnelles en santé, en particulier sur les dangers et les dérives du marché alternatif de la guérison et du bien-être, selon les derniers rapports de la MIVILUDES près de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique sont proposés : 1800 structures d'enseignement ou de formation sont jugés à risque 4000 psychothérapeutes autoproclamés n'ont suivi aucune formation et ne sont inscrits sur aucun registre 3000 médecins seraient en lien avec la mouvance sectaire et les dérives sectaires dans le domaine de la santé, représentant près de 40 pour 100 de l'ensemble des signalements reçus face à ces constats, il est nécessaire que soient menées des évaluations indépendantes et rigoureuses, des méthodes et des formations de pratiques de soins non conventionnels avant que soit envisagée, le développement de la médecine intégrative ne disposons pas à ce jour de de telles évaluations, nous devons faire preuve de prudence pour ces raisons je suis défavorable à ces deux amendements.

le budget de l'action 15, prévention des risques liés à l'environnement et à l'alimentation du programme 200 quinte et porté à 6 virgule 8 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de plus 28 % par rapport à 2000 22 et un budget bien supérieur aux années précédentes, depuis 2015, ce budget permet la mise en oeuvre de nombreux plans de santé publique, dont le programme national nutrition santé IV le fameux PNNS ce PNNS a pour objectif d'agir sur les comportements de la population en l'encourageant à se tourner vers une allocution une alimentation favorable à la santé tout en réduisant les inégalités sociales de santé à ce titre, il soutient et encourage le déploiement du nutriscore en France, mais également dans d'autres pays européens, le Nutri est un logo institutionnel en face avant des emballages faisant désormais l'objet d'une gouvernance transnationales coordonnées dans les 7 pays engagés en faveur du système toute évolution du Nutri Score est désormais gérée de manière conjointe avec les six autres pays et repose sur les travaux des comités de pilotage et scientifique de la gouvernance encadrés par ce mandat, le Nutriscore et donc un outil complémentaire aux autres mesures existantes ou futures, tels que les réglementations alimentaires, les autres labels de qualité ou encore de la filetage environnementale

ça n'était pas le SIDA, mais la maladie de Charcot, une demande de retrait, madame la sénatrice ou un avis défavorable, nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il est important de continuer les efforts de recherche sur la maladie de Charcot, mais néanmoins, nous apportons déjà des crédits qui sont jugés suffisants par les chercheurs pour pourvoir éventuellement continuer à avancer sur cette maladie, le plan France médecine génomique 2025 doit aussi permettre avancées dans la connaissance de la SLA et d'ouvrir la voie de meilleure prise en charge de cette pathologie et de sa recherche en développant une médecine de précision avec des thérapies ciblées pour toutes ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement sinon j'y serais défavorable. trente. à l'avant-veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, vous souhaitez augmenter les crédits en faveur de la prévention du VIH et des IST en diminuant les crédits du programme 183 des crédits sont déjà prévus sur le programme 204 pour le soutien aux actions tête de réseau intervenant dans le Champ de la santé sexuelle, j'ajoute que l'assurance maladie, contribue grandement à cet enjeu, via notamment le Fonds d'intervention régional les assurances de santé et de crédits alloués à l'Agence nationale de santé publique pour le financement des campagnes de prévention, l'action du gouvernement dans le cas de la feuille de route 2021 2024 de de clef, disons, de la stratégie nationale de santé sexuelle qui s'est donné notamment pour objectif de prix prioritaire de faire un pas décisif dans la diversification de l'accès au dépistage et aux outils de prévention afin de réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection par le VIH et les IST ou les hépatites et de poursuivre résolument l'information, la promotion et la formation à la santé sexuelle dans tous les milieux, à toutes les étapes de la vie pour agir en profondeur sur la perception de la santé sexuelle et favoriser la qualité de genre et la lutte contre les discriminations, des premières mesures concrètes ont d'ores et déjà pu être mis en oeuvre, notamment dans le cadre de la FSS pour 2022, possibilité d'accès sans prescription au dépistage du VIH du VIH dans les laboratoires de biologie médicale cette modalité de dépistage et d'ailleurs étendu aux IST, dans le cadre du Plfss 2023 pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement sinon j'y serais défavorable.

Madame Delmont sur la maraude, vous proposez de réduire les crédits relatifs à l'ANPE pour créer un nouveau programme d'accès aux soins, à la prévention des étrangers en situation irrégulière, je vous rappelle que, elle me donne droit à la prise en charge à 100 % des soins médicaux et hospitaliers, dans la limite des tarifs de la Sécurité sociale, les frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectuée dans le cadre de ses programmes de prévention sont en général pris en charge par l'AME ainsi les bénéficiaires de l'AME peuvent d'ores et déjà accédé aux consultations de prévention concernant les démarches d'aller vers la mesure 27 du Ségur de la santé qui vise à lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé a permis de renforcer le dispositif et des démarches d'aller vers notamment tourné vers les migrants 100 millions d'euros ont été mobilisés en 2021 à cet effet par ailleurs votre amendement suppose la création de l'aide médicale de santé publique qui souhaite recentrer la émeut sur les seuls soins urgents ou vitaux, je tiens à vous rappeler que remplacer la par un dispositif ne prenant en charge que les soins urgents les soins liés à la maternité et soins préventifs ne constitue pas une mesure efficace de maîtrise de la dépense, au contraire cela dégraderaient les finances publiques tout en engrangeant les services aux hospitalier pour ces raisons, je vous propose de retirer cet amendement, sinon je serais défavorable. Alors je crois que le 664 c'était l'écologie. C'était madame foncé Monge donc par votre amendement on vous proposez de créer un nouveau programme pour la transition énergétique et écologique du système de santé de 50 millions d'euros en 10 crédits, les crédits du programme 183. La transition écologique du système de santé est au coeur de la préoccupation du gouvernement, néanmoins, votre amendement est déjà satisfait par les différentes actions portées par le ministère de la prévention et de la santé, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir le retirer, à défaut, j'y serai défavorable. Et enfin, l'amendement 700 si vous permettez, je prends un petit peu plus de temps pour parler de Wallis et Futuna, donc par votre amendement, vous souhaitez renforcer les moyens affectés à la modernisation de l'offre de soins en diminuant les crédits du programme 183 il est important de rappeler que c'est à l'occasion de sa visite dans le Pacifique, les 21 et 22 février 2016 que le candidat devenu président de la République a pris l'engagement de l'installation d'une unité d'hémodialyse de proximité à Futuna afin d'éviter le transfert à Wallis des patients Futuniens souffrant d'insuffisance rénale, des financements pour créer une structure permettant d'accueillir les patients ont été débloqués, mais la mise en route des travaux a été retardé les travaux ont été entrepris depuis le mois de mai 2000 22 et devrait s'achever d'ici la fin de l'année, ainsi l'ouverture de ces structures d'hémodialyse sur l'île de Futuna permettra d'éviter les évacuations sanitaires vers l'île de Wallis pour ses patients dialysés pour ce qui concerne plus précisément les générateurs d'hémodialyse installé à Wallis, il s'agit de matériel de dernière génération, très performant et propriété de l'association pour la prévention et le traitement de l'insuffisance rénale ces générateurs permettent la prise en charge en toute sécurité des patients s'agissant enfin du transport des patients qui constitue une difficulté avérée à Wallis et Futuna, du fait de l'absence de moyens de transports publics ou de taxi, il est nécessaire d'y travailler plus largement avec l'assemblée territoriale du territoire sachant cependant que sur cette question qui n'est pas de sa seule compétence, l'Agence de santé met à disposition son ambulance pour la prise en charge des personnes à mobilité réduite devant se rendre à l'hôpital et peut ponctuellement véhiculé également des patients dialysés pour ces raisons je suis défavorable à votre amendement. Et je crois avoir répondu à tous les amendements merci madame la ministre, hé bien écoutez avant de mettre aux voix, j'ai de demandes d'explications de vote, tout d'abord Madame Jasmin. Merci madame la présidente, madame la Ministre, j'ai bien entendu les arguments et les éléments de langage que vous avez eu à propos de l'amendement que j'ai présenté, mais je crois qu'on ne vit pas dans le même monde parce qu'il y a eu encore aujourd'hui : manifestations dans les établissements publics de santé mentale, il y a de vrais problèmes de moyens, des moyens humains, des moyens matériels, il y a de grosses difficultés de prise en charge des patients donc vous avez peut-être de bonnes intentions, mais la réalité est là et les soignants, on n'en peuvent plus, alors il faudrait quand même mettent les moyens et là, j'ai proposé de flécher un budget spécifique pour la santé mentale afin que la prise en charge des patients soient réelles et c'est ce qui manque aujourd'hui, donc vous avez de bonnes intentions mais faudrait peut-être vous rapprocher des services spécifiques notamment sentimental et des des professionnels eux-mêmes pour qu'il puisse vous dire la réalité de leur quotidien, merci. Merci madame Jasmin Monsieur Savary. des choses à éclaircir pour voter des crédits pour faire de la recherche pour voir un peu ce qu'il est bon de ce qui n'est pas bon, néanmoins je suivrai le rapporteur qui m'a demandé de retirer l'amendement donc je retire l'amendement sur la médecine intégrative, par contre je maintiens bien sûr l'amendement sur la cryothérapie donc le le 254.

le problème urgent de Wallis, aujourd'hui il s'agit de problèmes de santé, de prise en charge ne vaut-il pas mieux conserver ses crédits pour permettre les soins sur l'île même au lieu de posséder à des évacuations d'urgence et de dernière minute vers la Nouvelle-Calédonie, de 450000 euros à l'échelle du budget, ce n'est rien du tout, et dès ce. Petit territoire à s'en sortir, c'est une question de santé publique aujourd'hui. Merci Monsieur Théophile Madame Cohen, vous avez la parole. Oui, c'est une explication de vote sur l'amendement 24 je pense. Que cet amendement ne prend pas du tout en compte la réalité de ce qu'elle a elle même et ça a été dit par plusieurs d'entre nous, ça constitue 0,5 % des dépenses de santé, et chaque année nous avons ce débat qui tire je trouve vers le bas et qui veut absolument raboter sur les crédits de l'AME et madame la ministre d'ailleurs dans son propos là l'a souligné, c'est une question de santé publique, c'est une question de de solidarité et c'est complètement contre-productif et je pense aussi que monsieur le rapporteur, vous n'avait pas connaissance de la situation réelle parce que être privé de titre de séjour n'empêche absolument pas d'être déclaré à la sécurité sociale et qui a, il ne peut Crisis terrible dans notre pays, il y a des pans entiers d'activités qui tiennent le coup grâce à des salariés qui sont sans papiers, pour la plupart, qui pèse, qui payent des cotisations sociales et qui sont super exploiter, d'ailleurs, le gouvernement est en train de réfléchir notamment un titre de séjour mais métiers en tension, donc il y a un vrai problème dans ce pays et il est complètement inhumain contreproductif et ne correspondant pas du tout

complètement cet amendement au niveau de mon goût. Merci madame madame Cohen Monsieur Bonhomme, vous avez la parole. Oui, madame la merci la présidente, Madame le Ministre, moi je voudrais juste revenir d'abord sur l'amendement 600 Weiss nutriscore plutôt l'éco-score je crois que le Nutri score à l'époque a été a été promu sans être rendu obligatoire parce que ils simplifient le message sur la valeur nutritionnelle du du produit, l'éco-score, c'est une autre démarche, et d'ailleurs une crise qu'on intègre les les aliments ultratransformés donc il ne faut pas tout confondre et je pense même qu'au contraire que le les Costco reviendrait nuire et est en train de lire une confusion qui serait dommageable je vous prends cet exemple dans l'éco-score, il est question de l'emballage plastique d'ailleurs de, de, d'apprendre que le rapporteur public du Conseil d'État a demandé l'annulation sur l'emballage plastique des fruits et légumes, mais, au demeurant, ça n'est pas en soi suffisante pour composer à me semble-t-il la notant ensuite je voudrais revenir Madame madame la présidence sur l'autre, l'amendement de Monsieur mouillé effectivement le bleu budgétaire concernant donc la carte vitale, la Madame le Ministre, le bleu budgétaire ne figure aucun crédit, je rappelle que l'été cet été au PLFR là l'amendement à la suite d'un avis de sagesse du Gouvernement avait été adopté, et donc là aujourd'hui vous faites mine de, de, de, de, d'avoir oublié les crédits alors même que ça deviendrait très simplement consacrer la volonté du Parlement de réaliser le chantier de la carte vitale numérique là le votre réponse sur les gars c'est parfaitement dilatoire si vous attendez l'IGAS alors que Didier en 2013, il a noté le problème que ça a été confirmé et accrédité par le rapport de notre collègue Nathalie Goulet que il y a eu d'autres rapports derrière qui ont conforté l'idée avec les auditions et là vous n'étiez que s'il faut attendre l'IGAS mais pourquoi pas le CNR et pourquoi pas aussi le commun sont citoyenne, qu'est ce qu'on attend simplement pour respecter mais la ministre et la volonté du Parlement et du Sénat, excusez-moi, par votre réponse, vous venez de piétiner la volonté du Sénat. Si cher collègue et pour terminer, la parole est à madame Gréaume. Oui, concernant le l'amendement 212 nous ne partons le contenu de l'amendement de nos collègues Les Républicains tous les chiffrages sérieux démontrer l'ineptie de ses discours sur les 40 milliards d'euros de fraude et les 8 millions de fausses cartes vitales en septembre 2022, l'assurance maladie a chiffré le surnombre de carte vitale 253250 Michalak, mes chers collègues, sommes-nous véritablement en train de débattre et de légiférer sur l'existence de 3200 sa cote carte en trop par rapport aux 51 millions d'assurés sociaux. Alors que les professionnels de santé ne souhaite pas devenir des policiers de la carte vitale que les assurés peuvent-elles également utiliser la carte vitale d'une autre personne en pharmacie que les ayants droit figureront toujours dans le dossier à midi et pas sur la carte, votre proposition de carte vitale biométrique est inutile, coûteuse, inefficace stigmatisante et obsolète, en effet, l'assurance maladie est lancé depuis fin 2022 une une carte vitale dans 8 départements, avec sa probable généralisation avec une application sécurisés sur téléphone, je vous rappelle que le rapport du Sénat de 2019 estimé que la mise en place de la carte Vitale biométrique nécessitera une dépense de 1 milliard d'euros et 20 ans pour renouveler l'ensemble des cartes, mes chers collègues, soyez cohérents avec votre opposition à la dépense publique et retirer votre amendement merci. par l'amendement 24 pour lequel j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe LR et le groupe socialiste, écologiste et républicain, je vous rappelle que. C'est un amendement présenté par monsieur le rapporteur de la commission des. Sinon, et que l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. le résultat nous avons. Votants : 343 exprimés 330 pour 199 contre 131 l'amendement est adopté. Et donc le 665

contre, abstention, il n'est pas adopté le 664. 2 avis défavorables, même avis même vote il n'est pas adopté,

donc l'amendement 212 qui a reçu un avis de la commission favorable et du gouvernement défavorable de procès de scrutin public dans les conditions fixées par l'article 55 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos.

Qui est contre cette-ci n'est pas adopté. Le 129 rectifié bis qui a reçu une sagesse de la Commission défavorable du gouvernement qui est pour. qui est pour. ça tient, il est adopté, le 130 rectifié bis qui a reçu une sagesse. De la commission, un avis défavorable du gouvernement qui est pour.

du gouvernement, donc c'est un avis défavorable de la commission ou sagesse alors ça ai de la Commission défavorable du gouvernement qui pour. Qui est contre qui s'abstient, il est adopté 2 avis défavorable sur le 706 qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté voilà alors peut être avant de compte. L'examen des amendements, il nous en reste 17 à examiner avant onze heures vingt donc je vous encourage est très bref dans vos argumentaires et dans vos explications de vote, sinon ça nous reporte comme vous avez compris. bien plus tard, le 685. Madame le président, madame la Ministre, mes chers collègues, un amendement qui porte une disposition assez simple, il s'est concernant les étudiants en dentaire, une aide à l'installation est prévu dans le cadre d'un contrat d'engagement de service public destiné aux étudiants et internes favorisant leur installation en zone sous-dotée depuis 2012 cet accompagnement est prévu pour les étudiants en dentaire. En contrepartie de cet engagement, les étudiants perçoivent une aide de 2000 euros et ils doivent à exercer leurs fonctions soit en une manière en libéral, soit en tant que salarié sur une durée égale au aux années correspondant au versement de l'aide, ou au minimum 2 années, il est proposé d'étendre ce le bénéfice de cet accompagnement des étudiants aux étudiants en dentaire dans le cadre d'une période de d'expérimental de deux 3 ans pour répondre aux besoins qu'il y a sur les territoires pour prendre la mesure de ses besoins, un exemple département que je connais bien, qui est la Nièvre pour vous dire les enjeux et la réponse qui ne sont pas le nombre, dans la Nièvre de de d'orthodontiste est inférieur à la la moitié de la moyenne nationale, un tiers des orthodontistes, en plus de 60 ans et 30 % de la population à plus de 60 ans, c'est dire les besoins de cette population liés au vieillissement, à des problématiques, comme les AVC, Alzheimer et autres maladies de ce genre, merci. Oui monsieur Joly, avis de la commission. avis de la commission. alors l'avis de la commission, les contrats d'engagement de service public sont financés par le Centre national de gestion de la fonction publique hospitalière sur des crédits d'assurance-maladie, la question de leur extension à d'autres étudiants que ceux des médecines ou notre d'odontologie peut difficilement être abordée dans le cadre de la mission santé donc demande de retrait ou avis défavorable. Merci, avis du gouvernement, Madame la Ministre. tous d'accord, vous proposer d'expérimenter le compte le CSP aux étudiants en orthophonie sur 3 ans, nous proposons un retrait si nous on avis défavorable, parce que l'idée de bien travailler sur toutes les professions paramédicales, et pas uniquement sur l'orthophonie, donc à un retrait ou un avis défavorable. Merci madame la ministre Madame Cohen pour explication de vote. avec le dispositif que vient de présenter mon collègue madame la mini-je vais en profiter pour attirer votre attention sur les orthophonistes et je pense que mes collègues présents qui vont visiter les hôpitaux les les établissements de santé seront tout à fait d'accord avec moi, quelles que soient les bancs de cette assemblée l'orthophonie manque cruellement de professionnels sur tous nos territoires c'est dramatique parce que un orthophoniste, une orthophoniste s'occupe de la prise en charge des troubles du langage, de la naissance pratiquement à jusqu'à la mort et il n'y a plus d'orthophonie suffisante sur le territoire aucune orthophoniste pour accompagner effectivement les enfants qui sont en difficultés de langage, mais j'attire votre attention, mes chers collègues, sur tous les trouble neurologique dégénératif dans les pas D'ailleurs, la maladie d'Alzheimer ou il n'y a pas d'orthophonistes et moi, pour avoir participé au Tour de France des hôpitaux avec mon groupe quand je demandais : vous n'avez pas difficultés avec les paramédicaux, la réponse était oui on manque de kiné mais les orthophonistes sont me disait rien et quand je demandais : mais qu'est-ce que vous faites sur les orthophonistes en neurologie, disait on se débrouille, hé ben on se débrouille pas parce que c'est la perte de chance pour les patientes et pour les patients, donc madame la mini-j'en profite pour vous dire : il faut absolument faire sauter le quota concernant les orthophonistes, c'est un numerus clausus déguisés, et aujourd'hui on a besoin d'orthophonistes, donc arrêtez de limiter leur nombre. je mets donc aux voix l'amendement 685 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est. Qui

madame la ministre hier, j'ai présenté cet amendement à votre collègue ministre de la culture qui m'a indiqué qu'elle s'engagerait à prendre attache avec vous pour que vous pour que celui-ci et toute votre bienveillance, donc je vais répéter rapidement ce que j'ai dit hier les associations de réduction des risques exerce depuis plusieurs décennies un travail indispensable auprès des usagers de drogue afin de limiter les atteintes à la santé individuelle et collective, ces associations sont par exemple présents dans de nombreux festivals ou concert pour sensibiliser le public sur les usages de drogues leur action permet de réduire le nombre d'overdoses d'identifier, de sensibiliser les, les, les usagers sur les produits les plus dangereux et de promouvoir des pratiques plus responsables, or cette présence essentielle est loin d'être garanties dans tous les événements à travers cet amendement, nous souhaitons pousser vers la généralisation de la présence de de ces associations en en milieu festif et culturel, bien souvent, ce sont les collectivités seuls qui accordent leurs subventions à ces associations, il est temps que l'État s'engage davantage. Merci monsieur dessus, avis de la commission, monsieur le rapporteur. à priori, vous êtes trompé d'amendements avis défavorable.

cet amendement vise à créer un fonds dédié à la recherche et à la prise en charge de l'endométriose cette maladie gynécologique chronique qui touche une femme sur 10 a un impact majeur sur la qualité de la vie des personnes atteintes avec un retentissement important sur leur vie personnelle, mais également professionnel et social pour autant les soins et la recherche reste aujourd'hui insuffisant en effet il faut 7 à 10 ans pour un diagnostic, voire parfois plus, il est urgent que notre pays accorde une attention renforcée aux événements de santé particulièrement marquant pour les femmes, alors que la stratégie nationale annoncée par le président de la République, malheureusement son calendrier ni budget spécifiques peinent à se matérialiser des avancées sur la prise en charge le diagnostic et la formation des professionnels de santé se font toujours attendre aussi l'amendement suggère d'allouer un budget spécifique pour accélérer la prise en charge d'un suivi adapté propre au corps féminin et propose une majoration des ouvertures de crédits à hauteur de 20 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement sur un nouveau programme recherche et prise en charge de l'endométriose. Si avis de la commission. Merci madame la présidente l'endométriose est certainement un enjeu de santé important l'amendement propose un budget spécifique pour accélérer la prise en charge d'un suivi adapté, mais on ne voit pas bien concrètement, quel type d'action devrait être financé par le nouveau programme proposé, ni si elle relève véritablement de la mission, je peux comprendre la volonté d'attirer l'attention du gouvernement sur ce point, mais la solution proposée ne me ne me paraît pas adaptée : demande de retrait ou avis défavorable. Madame la présidente, madame la sénatrice merci pour vous, en votre amendement que je considère plutôt comme un amendement d'appel donc le gouvernement à mettre un un avis de retrait ou un avis défavorable néanmoins prêté, permettez-moi de vous préciser que nous savons tous que l'enjeu De mettre sur la place publique, l'enjeu de l'endométriose ah, qui est une palette tologiques dont on parle trop peu, qui touche beaucoup de femmes, la stratégie nationale et se développe en 3 points : tout d'abord des enjeux sur la recherche avec 4 projets en cours de financement plus un programme d'équipement prioritaire de recherche de 20 millions d'euros sur 5 ans des enjeux de formation parce qu'on sait très bien que l'enjeu de la formation des étudiants en médecine est important pour pouvoir établir un diagnostic, il se fait depuis 2020 dès le 2ème cycle avec des programmes de formation interne et sur les sages-femmes est en cours, et aussi des programmes d'orientation prioritaire dans le cadre du dossier de formation continue et puis des tests salivaires permettront, nous l'espérons, de pouvoir faire des diagnostics assez précoce de cette pathologie, pour tous ces raisons nous émettons un avis de retrait ou défavorable sur votre amendement, néanmoins, nous sommes tous mobilisés pour avancer sur cette pathologie qui touche de nombreuses femmes. Merci madame vous maintenez votre amendement, il est maintenu, je le mets aux voix donc avec 2 avis défavorable qui est pour. qui est pour. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 686 Monsieur Jomier. Oui, madame la présidente, merci, donc cet amendement porte sur la situation de l'établissement français du sang qui nous préoccupe le FSE vit une période difficile avec une situation financière qui est structurellement déficitaire, c'est une situation qui dure depuis un certain nombre d'années d'ailleurs qui a amené à ce que des financements assurance maladie lui soit apportée de façon exceptionnelle, il y a plusieurs années, ces financements sont décroissant et se réduise à peu de choses maintenant l'EFS a mis en oeuvre une politique du coup de contention salariale, on va dire ça comme ça, les personnels ne sont plus suffisamment rémunéré, ils partent ailleurs les collectes sont réduites et la tension est vive sur les produits du sang et dérivés du sang, donc nous appelons le gouvernement à prendre la salle, la mesure de la gravité de la situation et à apporter les financements des sert à l'EFS au-delà d'autres réformes structurelles d'ailleurs qui sont nécessaires, c'est obligé de cet amendement. Oui, très rapidement, parce que c'est effectivement le même le même amendement le même esprit, simplement pour ajouter que notre amendement s'inscrit dans la continuité de l'Afrique. Colonisation du rapport d'information sur les médicaments de notre collègue député Pierre Dharréville afin d'assurer l'indépendance de la France en matière de médicaments dérivés et effectivement, il faut absolument préserver notre modèle français du don du sang donc madame la mini- je crois que les arguments ont été développés et nous vous encourageons à effectivement soutenir nos, nos amendements. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci madame la présidente, alors l'établissement français du sang n'est pas financé par ce programme, mais reçoit une subvention de l'assurance maladie qui vient compléter ses ressources propres auditionné la semaine dernière par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, son président, évoque un besoin de financement de l'ordre de 90 millions d'euros en 2023, tenant à l'impact de l'inflation à la nécessité des revalorisations salariales et à la baisse des ressources tirées de la fourniture de produits sanguins aux hôpitaux, je souhaite que le gouvernement puisse apporter des réponses sur les difficultés de cet établissement, qui joue un rôle fondamental dans notre système de santé souhaite avoir l'avis du gouvernement. Un avis défavorable sur ces deux amendements tout d'abord, permettez-moi de souligner le caractère exemplaire de l'AFS et de son personnel et de ses bénévoles pendant toute la crise sanitaire, je veux aussi rappeler c'est important l'attachement du gouvernement au modèle éthique c'est pourquoi le soutien financier apporté à l'EFS dans ses missions de collecte et d'approvisionnement s'est manifesté à plusieurs reprises les tarifs des produits sanguins, labile ont ainsi connu une augmentation de 3,3 % en 2021, les tests, les tarifs du plasma d'aphérèses utilisé comme matière première pour le fractionnement ont augmenté de 8 pour autant, le gouvernement est conscient du besoin aigu de financement de l'EFS notamment pour continuer d'attirer des professionnels de santé, l'EFS comme les autres établissements de santé, et lui aussi victime de la perte d'attractivité des métiers en santé, c'est la raison pour laquelle l'assurance maladie va en 2023, comme les années précédentes, contribuer à son financement par une dotation complémentaire de 25 millions d'euros enfin attentif aux tensions structurelles que rencontre l'établissement ainsi qu'à l'évolution de son activité comme de son environnement, le gouvernement va lancer très prochainement une mission des corps d'inspection pour évaluer le mode de financement de l'EFS et faire les propositions nécessaires à son adaptation. Mais merci, donc l'avis du gouvernement est un avis défavorable, le le l'avis de la commission pardon. Sagesse. Je me vois le six ah pardon Mesdames, pensez manche. Oui merci madame la présidente, je voulais soutenir ces ces amendements parce que, effectivement, il y a une vraie crise d'attractivité, Madame la Ministre, puisqu'il y a 200 à 300 postes vacants si si je ne m'abuse, et dans un de nos amendements, aussi, on rappelait que le l'EFS n'avait pas été bénéficiaire de la de la prime Ségur de 183 euros Net et que donc au delà des crédits que vous donnez, il serait temps qu'on aligne le EFS sur ça fait partie des oubliées du Ségur donc il est temps de remédier au CSA.

529 rectifié bis monsieur dessus, vous l'avez défendu alors ben avis de la commission défavorable gouvernement défavorable je mets aux voix l'529 qui pour.

Merci madame ah présidente cet amendement propose d'ouvrir une ligne budgétaire dédié au calcul de la prise en charge de tous les surcoûts des IVG pour les femmes et personnes concernées l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution, a été votée dernièrement à l'Assemblée nationale et reviendra sous peu au Sénat certains et certaines ici se sont opposés à la proposition de loi au motif principal qu'il valait mieux renforcer l'accès à l'IVG sur tout le territoire, hé bien, c'est parfait, nous allons leur donner l'occasion de voter notre amendement car n'empêche pas l'autre, au contraire, nous pouvons et nous devons reconnaître l'IVG comme un droit fondamental, tout en améliorant l'accès partout en France, nous nous réjouissons donc il y a une forte volonté de travailler sur l'amélioration de l'accès à l'IVG, car il est vrai que des restes à charge pèse sur les personnes concernées dans leur accès à l'IVG et peuvent effectivement être une entrave une difficulté un accès effectif à la à l'avortement, nous pensons notamment aux frais de transport, vous savez déjà que l'accès géographique un centre ou un personnel de soins performants des IVG n'est pas toujours évident en France d'ailleurs, suite aux fermetures des maternités et conséquemment des des centres d'orthogénie, vous savez aussi que la double clause de conscience des médecins, constitue à un frein supplémentaire, surtout dans des zones où il y a déjà peu de médecins ou d'hôpitaux bien en Angleterre, certains déplacements sont remboursés, nous pourrions nous en inspirer, et puis il y a les les possibles congé a déposé afin de pouvoir s'absenter du travail pour avorter, l'ensemble de ses frais concerne aussi les échographie de datation de vérification Post IVG qui peuvent être très variables à cause de la privatisation des soins, de nombreux hôpitaux publics n'ont pas les moyens de répondre à toutes les demandes et il n'est pas rare que de plus en plus de femmes se voient rediriger vers des cliniques privées, ce qui augmente de beaucoup les coûts donc cet amendement conclusion propose d'étudier les besoins en. Merci la hein, merci madame c'est mon avis de la commission

c'est pas la même chose quand même, il s'agit, il s'agit de et il fallait pas faire des scrutins publics, messieurs et mesdames, cet amendement propose l'instauration d'un congé spécial de 3 jours en cas de fausse couche, lequel pourrait bénéficier étant à la personne ayant fait une fausse couche jusqu'à son conjoint ou sa conjointe

sont dans un traumatisme, jamais reconnu et pris en charge, donc nous proposons d'ouvrir des crédits. C'est destiné à l'instauration et l'indemnisation d'un congé spécial de 3 jours. En cas de fausse couche. Merci, cher collègue,

Madame la Ministre, sur le scandale de l'empoisonnement au plomb par les industries, une campagne de dépistage a été menée contre le saturnisme dans le Pas-de-Calais après les révélations de pollution sur l'ancien site industriel de Metaleurop, 8 enfants sont atteints de saturnisme, Mai 68 sont concernés par le seuil de vigilance cette pollution des sols par le plomb qui concerne les sa commune limitrophe de cet ancien site industriel pose une meilleure anticipation des risques par les collectivités, avec les l'appui des moyens de l'État, les entreprises pollueuses doivent être mises à contribution pour la dépollution et pour l'Ademe Lisa Sion des victimes du saturnisme, de financer un nouveau programme pour l'indemnisation des victimes du saturnisme dotés de sacs 500000 euros merci. Madame la présidente, madame la sénatrice, vous le dites vous-même, c'est un amendement d'appel, je vais quand même apporter quelques précisions à à l'avis défavorable du gouvernement, les mesures de prises de prévention prises par les pouvoirs publics ont diminué, l'Exposition à ce métal de la population, les études disponibles confirment l'efficacité de la politique conduite par la baisse constante de la plombémie en population générale concernant la reconnaissance et la prise en charge de cette maladie particulièrement grave chez les enfants et les femmes enceintes, le saturnisme est pris en charge à 100 % par l'assurance maladie, enfin l'ARS peut être amené à contribuer au financement de certaines études en particulier aux études de santé ou la réalisation d'actes médicaux en mobilisant le fonds d'investissement régional, le cas échéant aussi votre amendement étant déjà satisfait, j'y suis donc défavorable. Je mets aux voix l'amendement 709 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui s'abstient, avis défavorables. Qui s'abstient, il n'est pas adopté de 708 madame Cohen. Oui, cet amendement d'appel vise à interpeller le gouvernement sur le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles subies par les étudiantes et les étudiants en médecine, notre groupe avait reçu l'association nationale des étudiants en médecine de France qui dresse un constat alarmant : Madame la Ministre, et qui souligne la détresse des internes, en effet, un quart des répondants ont été victimes d'humiliations ou de harcèlement sexuel, voire parfois d'une agression sexuelle ou d'un viol, ces violences s'exercent essentiellement sur le lieu de leur travail et le bien souvent par un supérieur hiérarchique, il donc extrêmement important d'apporter une réponse adéquate et d'empêcher effectivement ces violences de perdurer, surtout dans un contexte où vous le savez, toutes et tous, mes chers collègues, l'hôpital public public tient grâce à l'apport des internes, donc il constitue l'avenir notre système de santé notre amendement d'appel propose de créer un nouveau programme en faveur de la lutte. Contre la le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles dans le cas des études de santé doté donc de 200000 euros.

afin de de favoriser l'accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap par l'intervention de sage-femme auprès des femmes en situation de handicap accueillis en établissements médico-sociaux, je j'abrège selon le Fonds des Nations unies pour la population entre 40 et 68 % des jeunes femmes handicapées subissent des violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, 3 types d'actions doivent été déployé un suivi gynécologique adapté une information sur la vie affective et sexuelle et une information sur les violences faites aux femmes, pour les personnes accueillies dans les établissements, ainsi qu'une formation des professionnels de ces structures, voilà c'est une

pour les femmes, sur le plan gynécologique et que c'est des expérimentations sont notamment menées et j'ai pu le constater qu'en Normandie notamment cette exploitation et me c'est quelque chose d'important donc, merci pour votre amendement d'appel mais un retrait sinon un avis défavorable. Merci madame la ministre, je mets aux voix l'amendement 662 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. S'abstient, il n'est pas adopté, nous allons procéder au vote des crédits de la mission Santé figurant à l'état B je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'explique pis ration du délai limite je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission je mets aux voix les crédits de la mission qui est pour. qui est pour. S'abstient ils sont adoptés, j'appelle en discussion, l'article 46 bis et les amendements tendant à serrer un article additionnel qui sont rattachés pour leur examen au crédit de la mission. Santé

Bon, donc avis défavorable, je mets aux voix l'amendement de la commission des finances, qui a reçu un avis défavorable qui est pour. Qui est contre et s'abstient l'amendement est adopté le 909 Madame la Ministre, ça n'est pas un rédactionnelle. Un vrai rédactionnel madame la madame la présidente. Avis de la commission. Alors la, la commission n'a pas examiné cet amendement mais à titre personnel : avis favorable. Merci, alors je mets aux voix je mets aux voix l'amendement 909 du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission.

les comptes qui s'abstient, il est adopté. Après l'article 46 bis trois amendements qui font l'objet d'une discussion commune, monsieur le rapporteur monsieur Klinger. Merci madame la présidente, alors j'ai déjà présenté cet amendement que le Sénat a d'ailleurs voté en 2020, à l'initiative des 2 commissions finances et affaires sociales et sous une forme un peu différente, les 2 années précédentes, la France disposerait avec cet amendement, d'un dispositif de prise en charge des soins des étrangers, des étrangers en situation irrégulière, comparable à celui des autres pays européens. Merci, alors le suivant Madame Goulet, le 135. Oui, mais la présidente c'est un amendement de notre collègue, Véronique Louwagie, qui est rapporteur de ce budget à l'Assemblée nationale,

les soins dispensés, la lutte contre les tentatives de fraude, la lutte contre la fraude à l'aide médicale d'État, ce nouveau traitement automatisé de données permettrait de combler certaines lacunes observées dans le suivi des dépenses de l'AME cet amendement tient compte des observations formulées par la direction des affaires juridiques et ministères sociaux qui a été étudiée en 2021 donc il garantit l'anonymisation prévoit le renvoi au décret le renvoie à introduit une dérogation au secret médical, bref il remplit toutes les conditions qu'on lui avait demandé en 2021 pour être votée dans l'enthousiasme en 2022. Merci, cher collègue, le 676 Monsieur Jomier. Merci madame la présidente, en fait, en en le présentant, je vais réagir à l'amendement de Monsieur tout à l'heure, la présidente de la commission des affaires sociales, Catherine Deroche, disait la mission d'même au fond devrait être transmis à la mission Solidarité du budget, nous, nous proposons qu'elle soit transférée à l'assurance maladie, c'est l'assurance maladie qui maintenant, assure la prise en charge la définition des prestations et les remboursements et les ajuste en fonction de considérations de santé publique, la voix que prend la commission des finances, et malheureusement, semble-t-il, avec la commission des affaires sociales, qui est de vouloir définir un nouveau panier de soins dans le budget de l'État et les conditions d'accès à ce point panier de soins est une voix tout simplement se parce qu'en arrière plan, vous confondez un programme de santé publique, avec un programme de contrôle des migrations et ça n'est pas la même chose de faire de la santé publique et de faire du contrôle des migrations les deux sont légitimes, mais quand on a, on incite une confusion dans la législation, on a des dispositifs qui ne fonctionne pas, ce que vous avez voté en 2020 ne fonctionne pas, il était dans temps de transférer la M à l'assurance maladie, comme le demande l'Académie de médecine et on pourra refonder la discussion sur des bases saines. Merci Monsieur Jomier avis de la commission monsieur Klinger.

sur les lacunes du suivi des bénéficiaires de de l'AME j'indique par exemple dans mon rapport que l'effet des mesures prises en 2020 sur les nouvelles règles d'admission à la émeut et les mesures de lutte contre la fraude n'a pas été véritablement suivi, je ne suis pas certain que c'est là qu'une proviennent d'une insuffisance de données, les données sont nombreuses, tant dans les bases de l'assurance maladie que celle que dans celle de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, l'IGAS et l'IGF avait d'ailleurs pu y trouver des éléments particulièrement intéressant alors le développement est un peu long mais c'est une demande de retrait ou un avis défavorable concernant l'amendement du sénateur Jomier l'objectif poursuivi par l'amendement, à savoir la suppression du régime de la émeut et l'intégration des bénéficiaires à l'assurance maladie est en direction opposée à celui de la commission des finances, donc un avis défavorable. Merci madame la ministre, avis sur ces amendements. remplacer la AME par un dispositif ne prenant en charge que les soins urgents les soins liés à maternité les soins préventifs ne constitue pas une mesure efficace de maîtrise de dépenses quoi vous me présenter dans votre amendement au contraire cela dégraderait les finances publiques, tout en en argent à la fois les services hospitaliers, donc un avis défavorable sur l'amendement 135 vous proposer la mise en place d'un traitement automatisé de données à caractère personnel sur l'me poursuivent le dispositif et lutter contre la fraude, il s'agirait notamment de traiter de données relatives à la nationalité des demandeurs et bénéficiaires de l'AME ainsi que des données relatives aux pathologies soignées, cet amendement déjà proposé la dernière a fait l'objet d'une expertise juridique après analyse, nous ne pouvons pas envisager de mettre en oeuvre sous la responsabilité du ministère un tel traitement national comportant des données particulièrement sensibles à caractère personnel, donc un avis défavorable, et le dernier le 676, le gouvernement souhaite reste attaché à une séparation entre ce qui relève de la solidarité nationale et donc de la peau, comme l'allocation adulte handicapé ou la et ce qui relève du risque assurantiel encore majoritairement payées par les cotisations pour ces raisons, nous ne sommes pas favorables à cet amendement, donc un avis défavorable pour le 676. Merci madame la ministre, j'ai été saisi d'une demande de ah pardon Madame Cohen pour explication de vote. Oui, une explication de vote déjà on est intervenu au niveau de mon groupe, sur les différentes amendement qui sont portés par le rapporteur Klinger et qui vise à raboter sur la émeut mais je voudrais rajouter quelques quelques arguments supplémentaires, vous savez, mes chers collègues, à chaque fois que finalement on on mégote et que les soins sont tardifs en direction des personnes qui sont donc en situation irrégulière des étrangers et hé bien, finalement, ça coûte encore plus cher à la collectivité parce que c'est un problème de santé publique et plus les soins sont tardifs et plus ils sont coûteux, la 2ème chose quand même, et vous, vous vous devriez mais monsieur le rapporteur vous documenter davantage aujourd'hui 50 % des il existe 50 % de non recours à la M avec justement les risques qu'on peut imaginer sur la santé publique, donc vous essayez de brandir le drapeau de la peur alors que ce n'est pas conforme à la la, si la situation telle qu'elle existe et je le rappelle, notre groupe a proposé, a fait une proposition de loi pour que ce soit intégré à l'assurance maladie, c'est d'ailleurs ce que portent nos collègues du groupe socialiste et ce qui fait que nous avons le le même point de vue sur cette sur cette question, donc, ce que vous portez c'est très gras et c'est vrai que moi je déplore que, petit à petit, bien la commission des affaires sociales, dans sa majorité, hé bien, et gagné par cette thèse qui est plutôt une une thèse défendue par la droite extrême. Merci, alors j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe LR sur l'amendement vingt-cinq je vous rappelle que la vie de la, de l'du gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter Le scrutin est clos. Alors, résultat du vote sur l'amendement 25 votants, 343 exprimés 342 pour 211 contre 131 il est adopté. Alors, mais il fait tomber les 2 autres. Et nous allons passer au point suivant, à l'ordre du jour la parole est donnée à Monsieur Daniel Chassain pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci madame la présidente, concernant l'amendement 328 mon groupe souhaitait voter pour et je me suis abstenu

également pour une mise au point au sujet d'un vote. Oui, madame la présidente, je souhaite procéder donc à plusieurs rectifications la première porte sur le scrutin 81 ou mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe souhaité voter contre la seconde porte sur le scrutin 82 ou Loïc Hervé moi-même souhaitiez ont voté contre et Jean-Marie Vanlerenberghe souhaité s'abstenir je vous remercie. elles seront publiées au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique de scrutin. L'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission, plan de relance et de la mission investir pour la France de 2030 du projet de loi de finances pour 2023. La parole est à monsieur Jean-François Husson, rapporteur spécial de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial. La présidente, madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. La mission, plan de relance, c'est en voie d'extinction puisqu'elles n'ouvrent que des crédits de paiement d'un montant de 4 milliards 4, dont 3 milliards 6 sur le programme 362 écologie 0 milliards 4 sur le programme 363 compétitivité et 500 millions d'euros sur le 364 cohésion ces crédits de paiement permettront de poursuivre la réalisation de nombreux projets pluriannuels du programme 362 par exemple des actions de rénovation, réhabilitation d'investissement, voire de réalisation d'infrastructures, favorable à la transition écologique. Sur le programme 363 il s'agit en majorité d'actions relatives à leur relocalisation d'activités que 364 se limite désormais à des restes à payer sur les primes exceptionnelles alternance et sur certains dispositifs de soutien aux projets locaux. Les crédits réellement géré en 2022 sur la mission plan de relance sont assez différents de ceux votés dans la loi de finances initiale, car ils ont été accrues par des reports très élevé en crédits de paiement on est ainsi passé de 13 milliards d'euros en loi de finances initiale à 18 milliards en exécution en sens inverse des crédits ont aussi pu être transférés sur d'autres missions du budget général, la très grande taille des 3 programme et l'extrême diversité des dispositifs, si vous voulez bien quitter voilà ça ira mieux qu'ils permet au gestionnaire de programmes de procéder à des redéploiements en fonction du rythme d'avancement des projets ou des besoins sur venant en cours d'année cette gestion complexe Monsieur le Ministre, réduit, il faut le dire, la lisibilité de la gestion des crédits du plan de relance comme des missions qui contribue, en conséquence, le suivi des crédits est insuffisant, comme nous l'a dit la Cour des comptes dans le rapport qu'elle nous a remis au mois de mars dernier sur la mise en oeuvre des crédits, le plan de relance dans le cas où les crédits sont attribués aux bénéficiaires finaux. Par des opérateurs ou des entités publiques, autre que l'État, c'est le versement des crédits au tiers qui est retracée dans le système d'information Corus et non le versement aux bénéficiaires par ailleurs la décidé de justifier des dépenses au regard des jalons prévus par le plan de résilience européenne est une complexité supplémentaire, on peut constater, comme nous l'avions prévu un certain nombre de mesures portées par le plan de relance, qu'elles ne sont pas véritablement temporaire parce qu'elles avaient vocation à s'inscrire dans la durée, elles sont en conséquence, reprise par d'autres missions du budget général, notamment sur la mission Écologie développement et mobilités durables, un autre exemple malheureusement frappant est celui de la recherche duale, civile et militaire, ce programme traditionnellement porté par la mission recherche, enseignement supérieur, a été transféré pendant 2 ans sur la mission plan de relance sans augmentation de crédit et puis elle est revenue en 2023 sur sa mission d'origine, c'est avec de tels procédés, sans doute, que le gouvernement est parvenu à présenter un plan de relance de 100 milliards d'euros. De même, l'activité partielle qui avait été porté à la fois par la mission, plan d'urgence et par le programme 3 soixante-quatre cohésion de la présente mission sera à compter de 2023, financé par la mission Travail, emploi. Hé bien, on sort enfin de la confusion des genres que nous avions critiqué au total la mission plan de relance, a servi finalement de support de financement pour des mesures qui ne relevait pas de la relance de l'économie, au sortir de la crise de Covid 19 quant à la l'objectif de déploiement rapide, disons-le tout de suite, il n'a été du même que partiellement atteint le gouvernement espérait engager la totalité de cette somme dès 2021 et consommer les crédits de paiement progressivement finalement les engagements se sont poursuivies en 2022, malgré la reprise économique avec une telle lenteur que le taux d'exécution, un peu plus d'un mois avant la fin de cette année atteint à peine 55 % d'autorisations d'engagement et 45 % en crédits de paiement, c'est le ministre, il paraît clair que le gouvernement a une fois de plus constituer une réserve de budgétisation qu'il prévoit de reporter sur 2023. La Commission toute logique budgétaire vous proposera donc un amendement tendant à réduire les crédits du plan de relance d'un milliard d'euros car la mission plan de relance, créée en 2020 lors de la crise sanitaire n'a plus à être le support de nouveaux engagements en 2023 il sera suffisant de couvrir les engagements déjà pris, elle les crédits disponibles sont encore largement suffisant, la commission propose a donc l'adoption des clés de la mission, sous réserve bien sûr de l'adoption de son amendement, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général, la parole est à Thierry Mégnien, rapporteur spécial de la commission des finances. Madame la présidente de séance, monsieur le Ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. L'an dernier la mission Investissements d'avenir est devenue investir pour la France 2030, les crédits décidés au plan France 2030 il y ont été inscrits par amendement du gouvernement, sans en changer l'architecture, les 34 milliards d'euros du plan se sont donc ajoutés aux 20 milliards d'euros du programme d'investissements d'avenir, numéro 4 pays à 4 54 milliards d'euros, dédié donc au financement de l'innovation pour faire de la France, une terre d'excellence. En ayant intégré les crédits de France 2030 la mission prend une tout autre orientation qui est celle de soutenir l'ensemble du cycle de vie de l'innovation, jusqu'à son déploiement industriel en effet la logique porté par les pays à se situe en amont, elle est axée sur la recherche et la conception de l'innovation. Alors que celles qui anime, France 2030, se situe en aval, elle porte sur la mise en oeuvre de l'innovation et son industrialisation, rappelons que France 2030 cibles 3 priorités : celle de mieux vivre mieux produire, mieux comprendre notre monde qui renvoie à dix objectifs très concrets tels que faire émerger des réacteurs nucléaires de petite taille, devenir le leader de l'hydrogène, Vert ou encore produire 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici à 2030 et produire 20 biomédicaments contre les cancers et les maladies chroniques, notamment la mission qu'on prend donc aujourd'hui de programmes relevant du pays, à quatre et de France 2030 respectivement consacrés au financement des investissements stratégiques ainsi qu'au soutien des écosystèmes ensemble il rassemble 5 72 milliards d'euros en CP et également 3 programmes du pays, à trois, doté à hauteur de 369 5 millions d'euros en CP en 2023, ce pays a qui a été lancée en 2017 ne donne donc plus lieu à de nouvelles initiatives. Je retiendrai au titre des améliorations proposées en 2023 2 éléments : le 1er porte sur un changement méthodologique de calibrage des crédits de paiement qui a conduit à une réduction de 13 pour 100 des CP par rapport à la loi de finances initiale de 2022 ces crédits de paiements sont versés aux 4 opérateurs, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Ademe l'Agence nationale de la recherche BPIFrance et la Caisse des dépôts et consignations. La seconde amélioration concerne la gouvernance des projets, un contrôle inutile éré et mis en oeuvre, permettant ainsi d'émettre en cours de projet, des recommandations sur la prolongation ou l'arrêt du projet à l'issue des contrôles. Tout arrêt conduit au redéploiement de crédits autorisés en loi de finances rectificative si la finalité de la dépense ou la nature est modifié. J'en viens donc aux perspectives d'avenir, la mission affiche un objectif ambitieux 54 milliards d'euros pour soutenir l'innovation tout au long de la chaîne de valeur, de la recherche au déploiement je ne reviendrai pas sur les circonstances de l'intégration des crédits de France 2030 à la mission, certes, il fallait aller vite. Ce qui a amené quelques conséquences mais le constat cependant reste encourageant de nombreuses procédures de sélection ont déjà été lancés. Les auditions, nous ont démontré que le suivi des crédits par le SG pays et rigoureux. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant la gestion des crédits que la lisibilité de l'information donnée au Parlement afin qu'il exerce pleinement ses droits pendant l'examen du budget comme après l'urgence, à ses conséquences, ce qui a été gagné en rapidité de mise en oeuvre a été perdu en lisibilité, en effet, l'architecture actuelle de la mission est demeuré inchangé alors que la mission a pris une tout autre orientation elle n'offre pas la transparence, garantie par la LOLF l'an dernier, je vous alerter sur nos difficultés à suivre les crédits des différents pays à cette complexité s'est accrue avec l'ajout des crédits du plan de finances 2030 les intitulés des actions sont peu ou non thématisé, il est difficile d'identifier a priori la destination finale des crédits, il serait tellement plus simple de savoir que nous votons en 2023 pour la production de 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici à 2030, ou celle de 20 biomédicaments contre le cancer, plutôt que pour des innovations, je cite, je cite, titre d'une des actions, le gouvernement doit aller jusqu'au bout de sa logique : si la marque PIA disparaît au profit de celle de France 2030, cela doit se voir dans l'architecture de la mission, une organisation thématisé en 3 programmes correspondant aux 3 priorités du plan France 2030, permettraient de mieux identifier les politiques mises en oeuvre, compte tenu des facteurs d'amélioration constatée, la commission des finances vous propose donc d'adopter les crédits de la mission avec cependant les réserves suivante une amélioration attendue l'an prochain des mesures de la performance et la refonte thématisé de l'architecture de la mission à court terme, je vous remercie. Dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir,

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, comme certains l'ont rappelé la mission plan de relance, a été créée en réponse aux conséquences économiques de la crise sanitaire par la loi de finances initiale pour 2021, nous pouvons le reconnaître, le plan de relance historique pour redresser l'économie a bénéficié à bon nombre de particuliers, bon nombre d'entreprises et associations, collectivités ou administrations nous avons toutes et tous des exemples en tête dans le territoire respectif en somme, il s'agit d'investissement d'ampleur qui sont venus en aide à celles et ceux qui contribuent au développement économique, social et écologique de proximité à l'origine en 2021, ce sont 36,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 21,8 milliards d'euros en crédits de paiement qui ont été âprement acquis dans le cadre d'un plan de relance annoncé à 100 milliards d'euros, qui comprenait aussi d'importance d'importants allégements fiscaux et le volet européen qui prévoyait pour la France, quelque 40 milliards d'euros, le groupe RDSE a toujours salué ces politiques publiques ambitieuses qui répondait à des attentes tangible des forces vives depuis quelques temps. La guerre en Ukraine et le régime de sanctions cumulés avec les traces persistantes de la crise sanitaire ont en effet massif sur la conjoncture, ce qui pourrait rendre nécessaire un nouveau plan de relance, mais la lucidité budgétaire, a fortiori avec la remontée spectaculaire du coût de la dette publique nous malheureusement voir un idéal peu vraisemblable. Concernant les projections pour 2023, ce sont 4,4 milliards d'euros uniquement en crédits de paiement qui marque la continuité des prévisions de départ pour honorer les restes à payer, donc peu de surprises mais l'interrogation vient en effet de la gestion des crédits non consommés qui reporté, nous le savons, ce report s'explique en partie par l'envol des prix des matériaux qui rêve nettement l'investissement, tout est donc justifiée mais nous partageons le doute autour de la pertinence du transfert d'une partie de ses crédits vers d'autres missions du budget général de l'ordre de 1 milliard d'euros en autorisations d'engagement et 1 virgule 3 milliards d'euros en crédits de paiement en effet cela contribue à mettre de la confusion entre l'accompagnement financier qui relève du plan de relance, qui a été conçu sur une période donnée, et une mission qui relève de politiques publiques classique au sujet des programmes 362 sur l'écologie et 363 sur la compétitivité, si 364 sur la cohésion, nous n'avons pas d'observation supplémentaires au regard du fait qu'ils suivent des trajectoires ordinaire toutefois certains dispositifs liés à l'aménagement du territoire et au logement comme MaPrimeRénov'bouscule dans des missions de droit commun. Cela met en évidence une volonté d'inscrire dans la durée ces outils aux ambitions louables, mais nous pouvons effectivement regretter un manque d'évaluation sur l'efficacité avant prolongation s'agissant des crédits de la mission, France 2030, des crédits pour 2023 sont sensiblement plus importants, je me souviens de l'amendement adopté l'année dernière à l'Assemblée nationale, avec plus de 30 milliards en autorisations d'engagement un montant inédit pour un simple amendement budgétaire, ce que l'on appelait jusqu'à présent, les plans d'investissements d'avenir devrait conserver la même architecture avec une priorité donnée à la recherche et l'innovation. à l'heure de la réindustrialisation de territoire et de l'urgence climatique : le bon usage de ces crédits, plus que jamais nécessaire, faisons en sorte qu'il soit bien concentré sur les projets les plus innovants et non dispersée comme trop souvent, en somme, le groupe RDSE porte un regard favorable sur les crédits de ses missions avec vous l'avez compris les divers points de vigilance et je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Serge Babary pour le groupe Les Républicains

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits dédiés aux missions, plan de relance et investir pour la France 2030 la vocation du dispositif François Hollande c'était de prendre le relais des mesures de soutien aux entreprises mises en Oeuvres depuis mars 2020 mesures de soutien de masse, difficile à mettre en oeuvre, je regrette que certaines entreprises ont la situation été atypique emmener et en soient toujours exclus, ceci étant, la mission plan de relance, a été créé par la loi de finances pour 2021 afin d'aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, ce faisant, il s'agissait de passer de l'urgence à la relance économique, la mission alors été doté d'une enveloppe de 100 milliards d'euros, donc 40 milliards financés par l'Union européenne à engager d'ici fin 2022 avec 2 objectifs permettre à la France de retrouver son niveau d'activité d'avant crise et la préparer aux enjeux de demain, l'ensemble des autorisations de paiement ont bien été ouverte en 2021 et 2022 le présent projet de loi de finances Louvre donc sur cette mission que les crédits de paiement au mois de février dernier, nous étions tous réunis dans ce même hémicycle pour débattre de l'opportunité de l'efficacité des aides versées au titre du plan de relance, j'avais alerté Madame Pannier-Runacher, alors ministre délégué chargé de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les TPE et PME application trop stricte des critères complexité des dossiers, manque de transparence et d'individualisation, le meilleur exemple de cette complexité et l'annonce, il y a quelques jours d'un plan à venir pour la rénovation des bâtiments scolaires, cette annonce prend acte de l'échec du déploiement du plan France relance en ce domaine, alors que 950 millions d'euros était réservée à la rénovation des bâtiments publics notamment scolaire si je prends acte des efforts du gouvernement pour simplifier les démarches, je maintiens certaines de ses critiques, en particulier celles relatives à la complexité des dossiers et à l'absence de flexibilité, je souligne enfin l'importance d'améliorer le suivi et le contrôle de ces aides, le débat organisé au Sénat faisait suite au rapport du comité d'évaluation du plan France relance d'octobre 2021, ce rapport soulignait que si l'objectif de relance de l'investissement industriel en sortie de crise semblait atteint le court terme avait prévalu sur la transformation structurelle de l'industrie française, or depuis cette évaluation, rien, aucun nouveau rapport n'a été rendue publique la dernière action de ce comité, au mois de février dernier a consisté à lancé plusieurs appels à projets visant à évaluer le dispositif plan de relance, autrement dit des appels à projets pour évaluer d'autres appels à projets il est indisponible pensable disposer rapidement des évaluations des dispositifs passé afin d'en tirer tous les enseignements au mois d'octobre 2021 il y a un peu plus d'un an, le président de la République détailler les grandes ambitions de son nouveau plan d'investissement France 2030 destiné à préparer la France de demain en faisant émerger les champions industriels de demain un plan d'innovation et de réindustrialisation à 30 milliards d'euros sur 5 ans, complété par 4 milliards d'euros investis en fonds propres pour assurer l'indépendance stratégique du pays, la mission budgétaire investissements d'avenir, qui accueillait les fonds dévolus au plan d'investissements d'avenir PIA alors été transformée en une nouvelle mission investir pour la France de 2030, monsieur Bruno Lemaire là affirmé France 2030 et le pari d'une révolution de méthode basée à la fois sur l'agilité, la vitesse, la prise de risque et le pari de l'excellence, la semaine dernière dans une interview au journal Les Échos, monsieur Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement à afficher des objectifs extrêmement concret produire d'ici 2030, sur le territoire français, 2 millions de véhicules électriques des biomédicaments des avions bas-carbone des micros lanceurs spatiaux un robot sous-marin pouvant aller à 6000 mètres de profondeur ou encore former un 1000000 de personnes aux compétences de demain. On ne peut évidemment que souscrire à ces objectifs, même s'il semble bien lointain, alors que les Français sont confrontés à une pénurie de Doliprane et d'amoxicilline, envisager la fabrication en France de biomédicaments me semble un peu audacieux dans le présent projet de loi de finance la mission, France 2030 et doté de 262 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 6 milliards 9 en crédits de paiement de 18 novembre dernier madame la première ministre a annoncé son souhait d'accélérer le déploiement de ce dispositif, cette accélération traduit une prise de conscience de l'exécutif de la guerre commerciale en cours, une réponse aux mesures protectionnistes américaines contenues dans la loi sur la réduction de l'inflation, qui cherche à attirer les entreprises étrangères désireuses de réduire leur facture énergétique avec une enveloppe conséquente de 370 milliards de dollars une accélération qui s'inscrit dans un contexte de hausse probable des taux et de perte de liquidités, madame la première ministre, il s'est également engagé à simplifier les démarches des entreprises à simplifier le dispositif je souscris pleinement à ces objectifs d'investissements d'avenir et de renforcement de notre souveraineté industrielle, je regrette le manque de lisibilité de ces plans un peu fourre-tout qui se succèdent et conduisent et collectivités à endosser un rôle d'alerte de démarcheurs auprès des PME et TPE de leur territoire, il est important que, en dépit de ces différents plans, les entreprises puissent avoir un interlocuteur unique, enfin, je suis inquiet de la place de la France dans l'Europe quand l'Allemagne annonce elle aussi un plan d'aide massive susceptibles d'entraver la concurrence pour ces raisons, avec mes collègues du groupe Les Républicains nous voterons ces crédits mais nous resterons vigilants sur leur bonne emploi je vous remercie. Merci monsieur le président, la parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe, les indépendants.

Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La pandémie nous a cruellement rappelé à l'urgence du long terme et ce n'est pas le moindre des paradoxes qu'il n'aura fallu que quelques mois pour qu'un virus ne déstabilise le monde entier, mettant ainsi en exergue notre manque d'anticipation nos fragilités et nos trop forte dépendance, reconnaissons-le, aujourd'hui pendant de très nombreuses de trop nombreuses années voire des décennies nous avons négligé l'effort qui consiste à investir en portant une vision de long terme et privilégions la et en privilégiant la perspective de retour immédiat et de court-termisme la crise sanitaire nous a donc ramené à ce besoin de projection dans l'avenir de vision stratégique de long terme et c'est tout le sens que doit porter, France 2030 lancé il y a plus d'un an. Et qui vise donc à bâtir une stratégie d'investissement financier de développement économique et d'innovation scientifique et bien au-delà des cycles et ce bien au-delà des cycles électoraux cette projection dans le temps long, doit pouvoir rassembler au sein de notre assemblée de la gauche à la droite, pourvu qu'elle respecte la tradition française des plans quinquennaux, c'est donc dans cette longue tradition chère au général De Gaulle, qu'il est important d'inscrire ce programme France 2000 30 ans définition 3 axes de travail mieux produire, mieux vivre mieux comprendre et 10 objectifs ambitieux, le président de la République a présenté en octobre 2021 les priorités pour orienter le développement stratégique de la France sur les 10 prochaines années, cette projection répond aux attentes des investisseurs comme des industriels, les 54 milliards d'euros inscrits dans la mission si on avait ce Tir pour la France 2030 vise précisément à matérialiser ses ambitions, c'est considérable au regard de la plupart des autres missions, mais en l'occurrence c'est tout l'inverse des mots Talleyrand cantons sont qui disait : quand on on se regarde en sont console confond se compare on se désole, car la France demeure encore bien loin des objectifs de Lisbonne qui engage tous les pays européens à consacrer 3 % de leur PIB à la recherche et à l'innovation, la Chine, elle vient d'atteindre cet objectif, d'autres pays comme les États-Unis ou les ou l'Israël ou Israël ont compris depuis bien longtemps que c'était la condition même de leur développement et de leur souveraineté économique à venir, le succès de France 2030 ne résidera pas seulement dans les montants des crédits qui seront consacrés dans chaque loi de finances, l'efficacité de ce plan tient en grande partie à notre capacité à apporter des financements hoc aux entrepreneurs qui seront impliqués, les régions et, bien évidemment, ils prendront une étroite seront étroitement associés sur les territoires, je tiens à cet égard, a salué le rôle joué par le secrétaire général pour l'investissement, qui a fait naître beaucoup d'espoir, mais le bac malgré toute l'énergie déployée de nombreux hein entrepreneur sont impatients dans les files d'attente

mais nous ne devons pas les décevoir, le succès de France 2030 dépendra donc de l'de l'exécution des programmes de financement proposé aussi je rejoins le rapporteur de la commission des finances, sur la nécessité de renforcer les mesures de performance et de suivi de tels mécanismes l'éclairerais donc le travail parlementaire et nous ne pouvons qu'y être faut variable je pense toutefois qu'il serait intéressant également que la performance du dispositif soit aussi mesurée du du point de vue des entrepreneurs c'est-à-dire des usagers du mécanisme, cela nous permettrait de vérifier que nous ne ne retombons pas dans les travers des procédures administratives à rallonge on attendant de telles évolutions, notre groupe bien évidemment soutient le crédit de cette. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité territoire. Madame la présidente, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission, monsieur le Ministre, mes chers collègues, investir pour la France en 2030, quel grand sujet, je vous le dis, sans ambiguïté, je suis pour un plan d'investissement pour 2030 forts est conséquent, mais je déplore les orientations prises dans ce budget, quelle France veut ton pour 2030, le gouvernement se targue d'un plan France 2030, de soutien aux innovations écologiques, pourtant il est loin de répondre aux enjeux avion bas-carbone réacteurs nucléaires SMR, votre vision de l'avenir, ce sont les technologies qui sont censés répondre aux enjeux climatiques, vous faites fausse route si vous pensez que les gars technologique suffiront à répondre aux crises climatiques, on ne peut pas durablement épuiser les ressources de la planète, au-delà de leur capacité à se renouveler en 2030 dans l'Hexagone, selon Météo-France, le mercure pourrait régulièrement dépassé les 50 degrés les plus 1 virgule 5 degrés sont déjà jugées comme impossibles à obtenir par les scientifiques, il est donc urgent d'agir autrement, nous voulons accompagner à travers nos amendements sur cette mission à une véritable bifurcation du tissu économique français en donnant les moyens à la France de devenir la première économie de la transition en accompagnant les entreprises dans la durée pour transformer en profondeur leur modèle d'affaires, nous souhaitons conditionner les aides de la mission Investissements d'avenir au respect de véritable engagement écologique, bien sûr, cette mission, ils contribuent, dans certains domaines, je pense en particulier au crédit pour renforcer le potentiel de recherche et d'enseignement supérieur, avec ce plan, France 2030, comme c'était le cas pour le plan France relance les contreparties par contre ne sont pas au rendez-vous, les aides d'État doivent être conditionné à l'absence de versement de dividendes ou de licenciement non justifié pendant la crise, en effet, les entreprises du CAC 40 ont rémunérer leurs actionnaires à hauteur de 80 milliards d'euros au titre de l'exercice 2021 et risque de battre ce record au titre de l'exercice 2022, dans le même temps, elles ont annoncé 62500 suppressions d'emplois, dont 30000 en France, pourtant 100 % de ces entreprises du CAC 40 ont bénéficié d'aides d'État sans aucune contrepartie, quelle France voulait nous en 2030 des stratégies d'une ovation uniquement d'orienter sur la dématérialisation, la technologie et la domotique, il n'y a pas d'un côté les tenants de la modernisation et du progrès et de l'autre, les Amish qui s'y opposent, l'innovation, la création, la sobriété peuvent se conjuguer, mais votre approche à travers ce plan ignore trop cette exigence il est vrai que nous ne sommes pas convaincu que les métaverse ou les NFT, soit la meilleure cible d'investissements d'avenir pour la culture et pour l'humain d'une manière générale, il est vrai que nous défendons un modèle de consommation compatible avec la transition écologique et qu'il me semble indispensable de maintenir le soutien aux projets alimentaires territoriaux et aux solutions low-tech plutôt que de mettre tous les crédits pour les Start-Up de la Food tech de la grippe, souvent trop consommateur en énergie et en matières pour être généralisable. France 2030 devrait soutenir la recherche fortement sur la gestion de la ressource en eau, ainsi que la défense des écosystèmes sujet bouleversé par la crise climatique et pourtant essentielles à l'humanité, comme à la planète France 2030 devrait aussi travailler à la création d'un service public national de la dépendance, il devrait soutenir un véritable plan de reconstruction de l'hôpital public pour le préparer aux défis de demain, les conditions de travail, de l'ensemble des professionnels du soin et de l'accompagnement, continue à se dégrader pour sauver l'hôpital public, la réouverture de lits et services des dotations en fonctionnement suffisante, l'accès à la formation, l'amortissement de l'inflation, l'inflation pour 2022 2023 sont urgents, seuls, ces investissements permettront le choc d'attractivité tant attendu pour ces métiers nécessaires pour que notre service de santé publique redevienne un des plus performants au monde investir pour la France de 2030, c'est aussi donner les moyens à nos hôpitaux de poursuivent leurs recherches en s'appuyant sur des équipements performants voilà quelques pistes pour un plan d'avenir d'urgence à la fois social et écologique, chose que je ne retrouve pas dans cette mission, merci, merci. Si Monsieur seulement, la parole est à monsieur Jean Baptiste Lemoyne pour le groupe RDPI. madame la présidente, monsieur Ministre messieurs les rapporteurs, nous voilà réunis pour examiner ces crédits d'émission, plan de relance, France 2030, tout ça forme un continuum et que le plan d'urgence 140 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, 54 milliards d'euros respectivement c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent et ce sont des dépenses qui ont été de véritables investissements investissements en capital humain, vous évoquiez, monsieur le rapporteur, l'activité partielle, hé bien oui, il fallait garder ses talents, ses compétences pour relancer ensuite l'économie également investissement sur nos territoires, quand on regarde le plan de relance rejoint le collègue Gold, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on a vu autant de collectivités d'entreprises de ménages aidés, accompagnés avec ses crédits investissement tout simplement dans les technologies du futur, avec naturellement, France 2030 en quelques mots, parce que le temps est compté, le plan de relance ça quand même été une formidable révolution copernicienne au niveau européen, souvenons-nous des efforts qu'il a fallu déployer pour faire en sorte qu'on ait, c'est 750 milliards d'euros, que l'Europe puisse emprunter qu'on puisse avoir également des emprunts mutualiser et ça a permis 41 milliards d'euros qui vont abonder le plan de relance nationale ça a permis aussi d'aller, d'aller vite et fort, on évoquait les crédits engagés, je crois que c'est vrai que le périmètre de la mission un peu différente du périmètre du plan de relance en lui-même et sur le plan de relance, on est à 90 pour 100 de crédits engagés et d'ailleurs, il ne reste plus que 4,4 milliards d'euros de de CP cette année, vous le disiez monsieur rapporteur alors moi je me réjouis que un certain nombre d'actions soient reprises dans des missions de droit commun, ça monte, que l'État est de retour d'un certain nombre de politiques pour aménager du territoire avec le Fonds friche pour le tourisme, par exemple pour la rénovation des bâtiments publics et les résultats sont là, on le voit des trains de nuit, relancer la régénération des petites lignes ferroviaires, un chômage à 7,3 % vous le voyez, c'est vrai, c'est vrai, tant au niveau local qu'au niveau macro-au niveau national, quelques mots maintenant de France 2030,

à l'industrialisation comme vous le disiez, monsieur le rapporteur, et France 2030, c'est donc finalement voilà se rapprocher du futur avec 54 milliards d'euros d'investissement c'est massif, mais c'est nécessaire pour faire émerger des champions nationaux des technologies de demain avec une vraie boussole dans cette mission 10 objectifs 6 levier des indicateurs d'impact, hé bien tout ça, ça nous permet très clairement de préparer l'avenir et il y a d'ores et déjà 8,5 milliards d'euros qui sont investis à travers 1800 projets sélectionnés parmi les 50 appels à projets et puis tout ça innerve nos régions, nos territoires, un certain nombre de régions ont conventionnés, ce n'est pas de l'argent magique, monsieur le rapporteur, c'est magique parce qu'effectivement, la France va pouvoir aller de l'avant et je le vois également

et tout cela est possible aussi grâce à une maquette effectivement qui a été utilisé dans laquelle on a fait rentrer tout ça alors bon, c'est vrai, il faut peut-être la faire évoluer, mais c'est ce qui a permis d'être pragmatique voilà Action, réaction, je crois que c'est comme ça, hé bien, qu'on marque des points et en l'occurrence c'est la France qui marque des points, continuons dans ce sens-là en tous les cas, le groupe RDPI votera ces crédits pour toutes ces bonnes raisons. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur le président, Claude.

Madame. La présidente, monsieur le monsieur le Ministre, chers collègues, la mission plan de relance créée temporairement en 2021 avait vocation à permettre le déploiement de 100 milliards de crédits débloqués par le gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire pour relancer l'économie, si nous avions pu alors contesté le bien-fondé de la ventilation initiale des crédits ou le choix des actions à financer, comme par exemple et de façon un peu emblématique pour nous, la suppression de 10 milliards d'euros par an d'impôts de production, l'importance de cette mission budgétaire est désormais, il faut bien le dire bien réduite selon France Stratégie fin 2021 72 % de l'enveloppe de France relance avait été engagé 42 % décaisser et sa route la est estimé à 90 % cela a été dit, pour les crédits engagés en 2023 on s'engage donc sur ce qu'on pourrait appeler une queue de comète avec des cris de paiement de 4,4 milliards d'euros puisse un peu plus de 3 milliards d'ici fin 2025, ne serait-il pas pertinent, Monsieur le Ministre, du coup, de fondre pour le PLF 2024 cette mission avec la mission Investissements d'avenir, de manière générale, que de nombreuses mesures de France relance ont été au-delà du plan, ainsi en est-il de la part financée par le plan de relance de MaPrimeRénov'du Fonds, Free, c'est désormais intégré au fond Vert du bonus écologique de 7000 euros à destination des ménages modestes de la prime exceptionnelle à l'apprentissage des nouveaux appels à projets en faveur de la décarbonation de l'industrie troupeau tout projet qui se poursuivent aujourd'hui dans d'autres lignes budgétaires du point de vue de l'évaluation, les choses deviennent un peu difficile, il faut le dire, outre le fait que le comité d'évaluation, auquel nous participons, le rapporteur général je, je dois dire, nous devrions participer un peu plus, on va dire : il n'est plus présidée, vous le savez, après les nominations à d'autres fonctions des 2 animateurs précédents Benoît Coeuré et Laurence Boone et ce depuis l'été, nous n'avons plus de d'animateurs de ce de ce comité, nous le regrettons la crise ukrainienne et ses conséquences vont sans doute d'ailleurs rendre moins discernable à l'avenir dans leurs effets, les politiques de relance spécifiquement portée par ce plan, il y aura sans doute un mélange d'action très diverses, et il sera très difficile de, de savoir ce qui relève vraiment de l'action du plan de relance et ce qui relève d'autres d'autres politiques porté depuis les problèmes premières évaluations cependant, on en a quelques-unes dans un rapport chers collègue qui va vous être remis bientôt puisque nous avons pu travailler en visio avec l'ensemble des membres du comité pour pouvoir le sortir avant la fin de l'année, c'est en tout cas, ce qui nous avait été annoncé et donc, par exemple, les premières évaluations de MaPrimeRénov'en puisse cependant appelé à des modifications substantielles, l'impact de la mesure, notamment sur les passoires thermiques étant bien trop limité par rapport aux sommes engagées et donc il faut effectivement et cela a été proposé d'ailleurs dans le PLF modifier un petit peu les règles du jeu pour ce qui concerne la mission investir pour la France 2030 oh le pays à quatre intègre désormais le plan France 2030, on notera que, très logiquement, la gestion des autorisations d'engagement et des crédits de paiement demeure profondément divergentes, pour des raisons évidentes de lancement de programmes qui seront bien entendu déployés par des crédits dans le temps, notons cependant que les crédits relatifs aux pays à 3 de 2017 sont toujours déployés en 2023, alors on peut imaginer, c'était prévu pour fin 2020, mais on peut imaginer que les programmes ont pris du retard du fait de la crise sanitaire, bien entendu, mais vous nous direz : Monsieur le Ministre, au-delà de ces considérations générales, la commission des finances, par la voix de ses rapporteurs spéciaux Jean-François Husson et Thierry Mignon, aura à coeur évidemment d'analyser chaque année la progression, notamment de la consommation de ces crédits, tout à fait exceptionnel en faveur de l'innovation et de l'investissement industriel, pour ma part, je dois vous dire que je n'ai aucun doute sur le fait que la France se sera engagé ces crédits disponible de près de 54 milliards d'euros entre France 2030 et pays A4 dans des délais raisonnables, le seul vrai sujet en fait n'est pas l'engagement des crédits, je devrais pas le dire comme ça, étant président de la commission des des finances mais bon, encore une fois on sait dépenser de l'argent en France il y a pas trop de soucis, non, la question c'est : Soro nous finalement trouvé pousser les bons projets, c'est ça la question, saurons-nous également ce qu'on sait assez peu faire stopper rapidement tout projet qui n'tiennent n'irait pas ses promesses, Soro, nous serons-nous dans 10, 15 ans au rendez-vous des meilleures technologies innovantes, c'est en fait à cet horizon-là que nous pourrons juger de la qualité, notamment de la gouvernance mises en place, dont on attend beaucoup pour la gestion de ces crédits, en tout état de cause, ces programmes dont les pères en leur temps été je le rappelle, Alain Juppé et Michel Rocard, doivent être poursuivi et amplifié, si l'on veut que notre pays participe demain comme hier, à la compétition technologique que ce Live que se livrent les grandes puissances économiques, notre groupe votera donc les crédits de cette émission. Merci monsieur le président, la parole est à monsieur Pascal Savoldelli pour le groupe CRCE. Maître

Autrement dit, il reste 0 euros pour de nouveaux projets pour de nouveaux besoins. Si les dépenses encore prévues en 2023 à hauteur de 4 4 milliards la contribution de la mission à la croissance du pays apparaît toute relative. Et le risque de récession de l'activité économique pour 2023 est proportionnel au manque d'ambition de ce plan, le gouvernement a eu beau jeu de communiquer sur la rapidité du décaissement, la réalité est pourtant tout autre : si l'on compare les crédits consommés au crédit ouvert d'autres collègues l'ont exprimé trente-huit cinq pour portant 2021 ou en 2022 ou alors transféré à d'autres missions, les dépenses du plan de relance sont de nature hétérogène mais mais ont pour trait commun de se concentrer sur les mesures annoncées avant la présentation du plan mais non encore financées. Permettez-moi pour le groupe communiste de penser au Ségur de la santé au plan en faveur de la jeunesse ou bien à la location partielle de longue durée, le gouvernement a fait des les fonds de tiroirs des projets de Bercy et de quelques autres ministères pour définir et tenir un seul indicateur : la rapidité d'exécution du plan concrètement la démocratie parlementaire, votre 13 milliards d'euros pour la nommer le 22, hé bien le gouvernement ouvre unilatéralement 18 milliards donc l'empressement d'aujourd'hui engendre l'aéroport de demain, nous n'avons eu de cesse de vous alerter sur le caractère incertain des fonds européens et Monsieur le Ministre, mais votre gouvernement dans n'a pas tenu compte, à vous écouter, la France se voyaient promises le financement de 40 % de son plan de relance par les crédits européens finalement sont 2 milliards d'euros de subventions que notre pays n'aura pas explicatif l'exécutif s'employer à appliquer et là le doigt sur la couture l'agenda ultralibéral recommandées par les institutions européennes, on a vécu ce débat ici, la baisse des impôts dits de production, c'est fait, et voire même plus que promis la contre-réforme de l'assurance chômage, ça c'est fait, la contre-réforme des retraites, c'est en cours, donc vous êtes vraiment des bons élèves, ces mesures libérales ont fini par achever notre modèle social unique et par démanteler la protection sociale, annoncé à 100 milliards ce plan est amputé de 20 milliards d'euros de baisses d'impôts que vous consentez aux entreprises et qui pèseront chaque année chaque année sur nos finances publiques 80 milliards d'euros, donc, mais surtout les engagements pris n'ont pas été tenues où sont, par exemple, je vous pose la question : où sont passés les 6 milliards d'euros prévus dans le plan de relance pour le Ségur de la santé. Seulement un tiers ont été engagés, j'ai pas dit qu'il est avait rien de fait, soyez pas inquiets, un tiers ont été engagés au 31 août 2022 la promesse était belle, il y avait de quoi saliver, je cite, je vous cite : pas vous, votre gouvernement la modernisation nos nos établissements et à l'amélioration de la prise en charge des patients pour une transformation du modèle des Epad plus humanisé plus ouvert sur leur territoire et plus médicalisés et le véritable scandale sur Orpea n'y change rien, ces crédits ont disparu, il nous faut un engagement fort le plan un jeune une solution véritables fiertés du gouvernement est un gouffre financier. Et mériterait de s'appeler excusez-moi de le dire, un jeune hein précaire 10 milliards d'euros, soit 12,5 % des crédits du plan, c'est la somme qui devrait engager 10 milliards d'euros pour financer la subvention du patronat pour l'embauche d'apprentis ou encore l'aide à l'embauche de 4000 euros pour des jeunes de moins de 25 ans, les politiques d'emploi ne peuvent pas dépendre uniquement du patronat. On soutient la création d'emplois pérennes bien Méru un dernier point, le plan de soutien au secteur ferroviaire prévoyait des investissements pour 4 7 milliards d'euros, une somme indispensable dans tous les territoires pour un secteur indispensable à la décarbonation des mobilités, c'est plus de 4 milliards d'euros pour recapitaliser la SNCF et 650 millions d'euros Bienvenue destinés aux investissements dans les infrastructures de transport, il faudra donc ce plan de relance était insuffisant et nous voterons donc compte les crédits de cette mission, merci. La parole est à monsieur Michel Canevet pour le groupe Union centriste. a un monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, chers collègues, madame la présidente, alors c'est un sujet important que nous examinons bien entendu puisque les enveloppes sont conséquentes, mais je dois dire que nous avons parfois un peu de mal à nous y retrouver entre les plans d'investissement pour l'avenir entre les plans de relance entre les plans, France 2030 ou investir pour la France 2030, bref, il y a là un ensemble de de programmes qui, pour les béotiens sont difficiles à appréhender, en tous les cas, cela mérite quand même qu'il y ait une sorte de clarification qui permettrait aussi justement de bien clarifier les objectifs que l'on se fixe pour l'avenir de notre pays, et j'espère que c'est ce qui est contenu dans le plan France 2030 alors au niveau du groupe de l'Union centriste nous sommes particulièrement attachés à ce que il y a une bonne maîtrise des finances publiques et la problématique que nous voyons, c'est que ces programmes d'investissements qui ont été générés pour certains face à la crise que nous venons de connaître, je pense au plan de relance, fait que, hé bien quand on appréhende les Budgets ensuite amené à après après année si on intègre ces crédits que l'emploi considéré comme étant exceptionnel, on constate que finalement on arrive à une augmentation des dépenses de l'État, ce qui est particulièrement regrettable et donc, à notre sens, il faut que ces crédits restent exceptionnel et ne soit pas un truc intégré dans la trajectoire financière de la programmation pluriannuelle des finances publiques pour qu'on ait une trajectoire qui soit la plus vertueuse possible, en l'occurrence, que l'on puisse montrer une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement et que les dépenses d'investissement justement à préparer l'avenir et, bien entendu, nous en avons besoin alors l'Avantage que je vois sur ses programmes d'investissement c'est que on peut avoir une vision pluriannuelle et c'est vrai que pour ce qui concerne l'investissement, c'est essentiel, que l'on ne s'arrête pas à l'annualité budgétaire, mais qu'on puisse travailler sur la pluie réalité c'est l'avantage que j'y vois alors ce qu'il faut aussi, cela a été dit par les orateurs avant moi, c'est que nous puissions notamment bien évaluer les programmes qui seront de mise en oeuvre, on le voit, pour ce qui concerne par exemple le plan France rénovent qui est un point important pour permettre à chacun de nos concitoyens, en tout cas ceux qui en ont le le l'ambition de pouvoir réaliser des économies d'énergie et ainsi réduire l'empreinte carbone de notre pays,

des ambitions en la matière, donc il faut que l'on puisse montrer que ces programmes d'investissement ont effectivement un impact tout à fait pertinent alors sur les programmes de France 2030, monsieur le Ministre, bon je dois dire que un certain nombre de priorités ont été bien ciblés, il faut que tout cela puisse se mettre en oeuvre, je dirais de façon coordonnée, je pense par exemple à la question des bio-médicaments où l'on voit bien que l'on peut afficher une certaine ambition dans notre pays, mais les processus administratifs pour pouvoir aboutir à l'émergence de projets sont toujours extrêmement difficile, j'en connais un dans le Finistère par exemple ce que c'est et Marina qui, à partir de vers marins pour les greffons a mis beaucoup de temps à pouvoir concrétiser la validation de de son produit, qui pourtant était utilisé à l'étranger, on voit bien que nous avons encore des circuits administratifs dans notre pays qui sont particulièrement lourd, particulièrement difficile et qui empêche l'émergence d'un certain nombre de projets pourtant important dans ce projet, France 2030 a été aussi évoquée tout-à-l'heure par mes collègues, l'objectif de 2 millions de véhicules de production de 2 millions de véhicules électriques dans notre pays, il faut qu'on soit attentif effectivement à ce que cette ambition que légitimement peut afficher de produire des véhicules décarbonés hé bien que les dispositifs que l'on maison en place dans notre pays aille effectivement pour l'émergence des produits fabriqués en France, la prime aux primes de passage aux véhicules électriques, il faut qu'on s'attache à ce que ces ces primes soient effectivement versées pour des véhicules effectivement ou en Europe mais pas des produits qui viennent forcément de l'étranger qui vont contribuer à accroître la balance le déficit de la balance commerciale qui ait des gens extrêmement lourd, hélas, Monsieur le Ministre et ça monte, cela montre bien les efforts que nous avons encore à faire pour revenir à, à un meilleur équilibre ce plan France 2030 évoque aussi mais de façon extrêmement comme d'ailleurs les programmes antérieur, une ambition pour la mer, je dirais, pour que la France affirme sa vocation maritime, c'est extrêmement important parce que la France possède le 2ème espace maritime le plus étendu, le plus vaste au monde on a parfois l'impression que nous n'avons pas une ambition assez forte en la matière, je veux dire par là que bah, nous soutenons par exemple, l'aviation, le vraiment de l'aviation bas-carbone nous devrions aussi Monsieur le Ministre, soutenir le développement des navires bas-carbone c'est important parce qu'on voit bien que l'essentiel des flux de marchandises se passe par la voie maritime, donc il est important que l'on puisse agir en ce sens, voilà le groupe de l'Union centriste bien entendu adoptera ces crédits. Merci, cher collègue. Alors la parole est maintenant à monsieur Roland Lescure Ministre délégué chargé de l'industrie. Merci madame la présidente, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les sénateurs. En début du mandat précédent, le gouvernement avait clairement adopté une politique qui visait à réindustrialiser la France et à favoriser l'innovation avec des baisses d'impôts avec une stabilité des des crédits destinés à mobiliser l'innovation avec la simplification des règles présente dans la voie pas que la loi ASAP et cetera, et cetera, mais il faut bien reconnaître que la crise du Covid inédite évidemment dans son ampleur, a aussi constitué une opportunité inédite pour mettre en place à prendre, relance lui également tout aussi inédit je parle évidemment du plan France relance dont nous discutons aujourd'hui de la fin ou presque des crédits des moyens sans précédent, avec 100 milliards d'euros, dont je souhaite rassurer le sénateur Savoldelli 40 milliards donneront bien lieu inversement par l'Union européenne, qui a déjà versé plus de 5 milliards en 2021 plus de 7 en 2022 plus de 13 en 2023 et ça va continuer, avec des priorités claires la transition écologique, la compétitivité et la cohésion nationale, alors que la mission relance arrive à son terme le bilan, je pense que ça a été quasi unanimement reconnu sur ces bancs, et d'ores et déjà extrêmement positif, les retours des acteurs économiques sont. Unanime 35 milliards ont été engagés pour soutenir l'industrie qui m'cher 30 milliards pour la transition écologique avec ça a été dit par le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne 70 % d'engagement en décembre 2021 et 90 % en août 2022, c'est tout bonnement exceptionnelle, j'entends que du coup l'efficacité a primé et que parfois, notamment sur des des outils de suivi ça été mentionné par le monsieur le rapporteur général de Corus a été parfois un peu difficile de retrouver nos petits mais je pense que l'urgence était extrêmement importante à l'époque, on se souvient d'une récession historique qui a affecté la France et le reste du monde et je pense qu'on peut tous être collectivement assez fier du fait que la France est sortie de cette ornière historique avec une dynamique sans précédent et que c'est en grande partie grâce à France relance qu'elle le doit quelques réalisations très concrètes : la rénovation énergétique des bâtiments, ça a été dit perfectible, mais elle a été quand même lancé des infrastructures, la mobilité verte, la biodiversité, la transition du modèle agricole je souhaiterais rassurer le président barbarie qui l'évoquait tout à l'heure le rapatriement du paracétamol, qui a lui aussi été en partie favorisés par France 2030, bref des exemples très concrets de résultats très concrets d'engagement très concret que vous avez les années précédentes, mesdames et messieurs les sénateurs voter. Les résultats sont flagrants aussi d'un point de vue macro-économique, je vous le rappelle, dès la fin 2021 l'activité française avait retrouvé son niveau qui prévalait avant la crise, l'emploi a lui suivi dès la mi-2021 et l'emploi industriel qui m'est cher, et lui aussi aujourd'hui au-dessus en France de ce qu'il était avant la crise, on a connu une reprise en V en France qu'on n'avait jamais connue auparavant, là encore, soyons-en fiers je rassure l'ensemble des sénateurs qui se sont interrogées sur l'avenir du rapport Kev écoeuré oui Benoît qui Coeuré a été nommé président de l'Autorité de la la concurrence mais les travaux de la commission continue, elles ont déjà conduit à l'évaluation macro-économique du plan France relance et de 5 priorités, il en reste une dizaine qui lui avait été conseillé, elles seront également évaluée. Et puis, pour reprendre l'expression du président rénale, on est dans la queue de la comète du plan de France relance mais on peut dire quand même que cette comète, elle a bien briller, elle a été très efficace et nous pouvons tous je pense en être fier, pour autant, ça a été dit sur ces bancs, nous arrivons à la fin de ce programme et il est temps de passer, j'allais dire à autre chose face à des défis qui sont extrêmement nombreux, la crise énergétique, on en passe, on en parlera pas ici ce soir, mais elle est là et bien là, celle dont on parle aujourd'hui, je pense, c'est l'accélération technologique qui a lieu partout dans le monde et qui fait que des grandes zones économiques comme les États-Unis, la Chine et l'Asie en général ne nous attend pas, pour continuer à innover pour investir de manière massive dans la transition écologique, j'allais dire en ce qui concerne les Etats-Unis, il était temps, et donc nous devons répondre à ce défi technologique majeur, un des défis auxquels nous faisons face auquel s'ajoute un 2ème défi tout aussi important, la fin de l'argent facile, la fin de la surabondance de liquidités qui fait que les taux d'intérêt sont en train de monter que le financement est plus difficile, notamment pour les acteurs émergents pour les acteurs innovants, pardon, France 2030, qui a été engagé il y a un an par le président de la République, quasiment jour pour jour, c'était en octobre, qui vise, ça a été bien dit par certains d'entre vous à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation à positionner la France non pas seulement comme un acteur, mais bien comme un leader du monde de demain pour répondre aux défis écologiques démographiques, économiques, industriels et sociaux et je rassure, de ce fait, le sénateur Salmon, les investissements de France 2030 sont évidemment conditionnée à des progrès majeurs sur toutes ses dimensions, ça fait partie je pense de la beauté de la chose, France 2030, c'est à la fois une action ciblée sur des priorités : pas de saupoudrage extrêmement structuré le sénateur Lemoine nous les a rappelés organisé en ascendant pour ne pas mentionner le terme de bottes aux que le rapporteur nous a je je dirais justement reprocher en attendant en partant des projets pour laisser tout son Champ à la créativité, à l'initiative et à l'esprit d'entreprise, je rajoute pour compléter la description de ce programme, je vous le rappelle, que nous investissons toujours systématiquement en parallèle avec des investissements privés, nous ne sommes pas dans le gaspillage de l'de l'argent public, mais bien dans l'accompagnement d'investissements innovants qui vise à accompagner les acteurs privés dans le développement de la France de demain, les cibles sont ambitieux, ça a été dit également en montant 54 milliards d'euros, investir sur 5 ans, c'est 5 fois plus que les 2ème et 3ème programme des investissements d'avenir, en soutien aux petits acteurs, je sais que vous y êtes extrêmement sensible 50 % des crédits seront destinés à des petites entreprises, des entreprises de taille intermédiaire innovantes et en ambition écologique avec 50 % qui seront destinés à des projets bas-carbone ou de décarbonation et au total 0 nuisibles à l'environnement. Tous les projets sont évalués à l'aune de critères extrêmement précis, je les mentionne rapidement parce qu'ils font l'objet d'amendements de la part d'un certain nombre de sénateurs sur ces bancs ce soir autour de l'innovation, des effets d'entraînement territoriaux, je sais que vous y êtes sensible aux emplois créés à la décarbonation à l'autonomie stratégique et la souveraineté au capital Hurme au Leadership et à la mixité, notamment l'égalité femmes-hommes se cause qui m'est particulièrement chère à l'issue de la semaine de l'industrie, qui nous a beaucoup occupé sur cette cause importante de ce fait, il ne nous semble pas nécessaire de rajouter des programmes particuliers sur chacun de ces critères, ce qui expliquera notre avis défavorable à certains amendements que vous avez déposé

plus de 8 milliards engagés en un an, d'ici la fin 2022, on sera sans doute à 10 milliards avec plus de 1700 projets soutenus et 1300 entreprises sur 5300 entreprises c'est important, plus de 60 pour 100 de PME et de Start-Up nous remplissons l'objectif et, au-delà, d'avoir un soutien extrêmement précis pour les petites entreprises et dans les territoires, puisque près de 60 % des fonds alloués le sont hors d'Île-de-France, vous nous avez remontées et d'autres l'ont fait avant vous, des difficultés qui nous conduisent à adapter le programme notamment le foisonnement des dispositifs le rythme d'instruction souvent un peu trop long, ça a été dit, ici la complexité et le poids des procédures, le risque de rater la date d'un appel à projets, souvent un peu couperet, nous agissons pour simplifier tout ça nous accompagnement en nous accompagnons pardon les acteurs en proximité avec les services de l'État avec les opérateurs, les chambres de commerce et d'industrie nous Ziad également les pôles de compétitivité, et caetera, nous suivons les délais au plus haut niveau, j'en fais une de mes priorités, je suis membre des comités de depuis pilotage ministériel de France 2030 en tout cas, 9 d'entre eux sur 14 et ce sujet des délais et systématiquement mentionné et évaluer l'accessibilité des appels à projets nous est aussi extrêmement cher tous les appels à projets sont disponibles et de manière extrêmement lisible sur le site gouvernement les sénateurs et aussi les projets qu'il souhaite porter dans leur territoire, allez le voir ce site était extrêmement bien fait, nous avons d'ores et déjà des avancées concrètes que je ne vais pas détailler, mais sur la décarbonation sur les réacteurs sur les giga factories nous finançons des pré-séries de nouvelles machines agricoles, bref, France 2030, ça marche, nous devons accélérer une trentaine d'universités ont été soutenues partout sur le territoire, notamment en Corse et dans les outre-mer pour finir : notre objectif est extrêmement clair : nous voulons préparer notre avenir, nous voulons renforcer nos atouts réduire nos faiblesses, donner de la visibilité aux porteurs de projets à faire le choix du meilleur parce que nous faisons le choix de la responsabilité budgétaire mais aussi de l'excellence, France 2030, est un programme sélectif et le restera, je vous remercie. Je vous rappelle que pour ses missions, la conférence des présidents a fixé la durée maximale de la discussion à une heure quarante-cinq en conséquence, si nous n'avions pas terminé l'examen de cette mission à une celle-ci se poursuivraient à la fin d'émission de la semaine et nous allons entamer donc cette discussion par 2 amendements qui font le l'objet d'une discussion commune le premier, le vingt-sept, monsieur le rapporteur spécial au nom de la commission des finances. Oui, qui consiste à proposer de une mesure d'économie, puisque il reste. Un peu d'argent, et quand je dis un peu suffisamment en tous les cas, je propose de sincériser le dispositif, on a en, comment dirais-je, en enlevant un milliard d'euros, et en le prélevant sur un certain nombre de programmes compétitivité cohésion, voilà ce qui permet, il y a en plus, il y a de la réserve, je l'ai dit dans mon dans mon propos lors de la discussion générale, donc ça a le mérite d'être parfaitement clair et de ne nuire en rien aux besoins des autorisations d'engagement, d'ores et déjà déployés. Merci, monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, c'est un aveu. Excusez-moi, monsieur le Ministre, on est en discussion commune. à l'heure, on va prendre le 206 avant de vous demander votre avis, excusez-moi, monsieur le Ministre.

par le prélèvement de 262 millions d'euros sur l'action souveraineté technologique et résilience du programme, compétitivité, la création d'un pôle public du médicament, alors que les ruptures de stock de médicaments explosent avec récemment des médicaments très utilisés, comme le Gaviscon, traitement contre les brûlures d'estomac ou le Doliprane, désormais ce sont les stocks d'amoxicilline qui sont menacés, l'Amoxicilline est présent dans près de 80 % des antibiotiques pédiatrique et pourrait devenir une denrée rare, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les formes dites buvable d'amoxicilline utilisés dans le cas de traitements pédiatriques connaissent de fortes tensions d'approvisionnement qui sont prévus, et là, jusqu'en mars 2023 cet antibiotique s'ajoutent aux 2160 médicaments concernés par des ruptures de stock, face à cette situation, il y a urgence pour notre pays de recouvrer notre souveraineté sanitaire de ne plus dépendre des industriels du médicament qui ont délocalisé leur production en Asie il y a urgence à recréer une production en France des molécules essentielles pour éviter les ruptures de traitement de nos concitoyennes et concitoyens, notre groupe avait déposé une proposition de loi en 2020 en ce sens et nous estimons indispensable de mettre en place et de production publique de médicaments et des produits médicaux, comme vous le savez l'Agence générale des équipements et produits de santé, la JEP, ce produit des médicaments et des molécules pour les hôpitaux, la pharmacie des en produit également pour nos militaires en leur donnant plus de moyens, on pourrait franchir une première étape dans cette production de molécules essentielles, donc nous avons toutes et tous vécu les conséquences de la crise de la Covid 19 il faut en tirer ensemble les enseignements car la pénurie qui frappe un certain nombre d'antibiotiques, crise d'ouvrir sur une crise de la santé absolument majeur telle et le sens Merci madame la présidente, créé de toutes pièces et donc sans autorisation d'engagement des crédits de paiement mais ça a été abordé par d'autres, la question. De la souveraineté en tous les cas de de la reconquête de la souveraineté autour du médicament, produit en France.

parce que vous tablez sur le fait que d'ici la fin de l'année, l'ensemble des autres, des autorisations d'engagement ne serait pas complété, je souhaite être à la fois plus optimiste et plus volontariste que vous nous avons montré jusqu'à présent, nous savons engager les crédits à hauteur extrêmement ambitieuse, nous avons prolongé, je pense, la date limite d'engagement au 23 au 26 décembre 26 décembre et je souhaite véritablement et je dois vous avouer que ça crée une certaine incitation pour les administrations, à ce que l'ensemble des autorisations d'engagement de France relance puisse être engagée et au cas où je serai dans le vrai votre amendement nous conduirait à avoir un milliard en moins l'année prochaine qui risqueraient de déséquilibrer le budget, donc je le regretterai, donc c'est un avis défavorable sur l'amendement du rapporteur général et sinon une demande de retrait pour le soir. Merci, monsieur le Ministre, alors si y'explications de vote Madame Cohen. Oui, quelques secondes, monsieur le mini je veux quand même attirer votre attention parce que l'intervention que j'ai fait et et l'amendement que j'ai défendue par rapport à un pôle public du médicament englobe la la la production, la diffusion mais vous interpelle, vous également en tant que ministre qui vous occuper de la réindustrialisation du pays parce que à chaque fois que nous ne pouvons au niveau de mon groupe, hé bien, on pose la question au niveau du ministre de la Santé, on vous pose la question, et c'est toujours une fin de non-recevoir, or on est dans l'urgence concernant la production de médicaments et ça fait partie d'une de vos prérogatives donc monsieur le mini j'attire fortement votre attention et je vous appelle à être attentifs à notre proposition. Merci madame Cohen pas d'autre explications de vote, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe LR sur l'amendement 27 je vous rappelle que l'avis du Gouvernement est défavorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

personne ne demande à voter, le scrutin est clos. Alors le résultat du vote sur l'amendement numéro 27 Votants 343 exprimés 279 pour 243 contre 36 il était adopté. Et donc l'amendement 206 tomber le 156 rectifié bis, c'est monsieur. Savoldelli qu'il défend, il est défendu. Ah pardon Madame à Madame Jourda, pardon, excusez-moi.

alors Monsieur le Ministre, je vous prends au mot, vous avez dit freins se relance, ça marche, j'espère en tout cas que ça marchera pour cet amendement transpartisan lié à un fonds de dépollution et qui augmente le montant des crédits de paiement du programme écologie de la mission, plan de relance de 64 millions 400 1000 euros, pourquoi, parce qu'à l'aune de 2023, le plan présenté prévoit de n'ouvrir que 10 millions 600 1000 euros pour le fonds recyclage friche enveloppe ancien site industriel à responsable défaillant dispositif sous responsabilité de l'Ademe, page 33 du bleu budgétaire, les membres de la commission d'enquête sénatoriale sur les problèmes sanitaires et écologiques liés aux pollutions des sols qui ont accueilli des activités industrielles ou minières, estiment unanimement à ce jour que ces crédits sont largement insuffisants au regard des besoins à la matière et des coûts inhérents à la dépollution et à son suivi partie de ping-pong, plan de relance au fond Vert, tout ceci est bien confus et il est temps de sortir des amalgames, le rapport de notre commission d'enquête éclair sur le sujet 75 millions d'euros annuels sont nécessaires pour abonder un fonds dédié au financement de la réhabilitation des sites et sols pollués comprenant bien entendu donc les sites orphelins malheureusement balayé à l'Assemblée nationale, il y a 2 ans, cet amendement, mes chers collègues, nous l'avons déjà adopté au Sénat il y a 2 ans, ne baissons pas les bras, inscrivant notre volonté de sortir de la situation à l'adoptant gagées sur le programme Compétitivité, il explique : un bon geste, Monsieur le Ministre, celui de lever le gage je compte sur vous et vous remercie. Merci, cher collègue, monsieur le rapporteur spécial à vide, la commission. Donc un, un amendement qui propose d'abonder le le Fonds friche à hauteur de 64 millions d'euros je rappelle juste à notre collègue en 2023 et a passionné Comme d'ailleurs d'autres mesures du plan de relance et repris par la mission Écologie Mobilité et Développement durable, donc on ne va pas, je pense qu'il faut éviter de doubler les dispositifs, il n'est donc pas souhaitable de le financer également également sur le plan de relance qui est en voie d'extinction comme je l'ai dit tout à l'heure donc une demande de retrait, même si le la cause est noble et je pense qu'il faut la porter, mais sur le bon programme de la mission Écologie. Merci, monsieur le Ministre. Non, mais ma vie, je rajouterais juste que le Fonds Vert qui est porté, vous l'avez dit dans la mission Écologie et être abondé à hauteur de 300 millions d'euros et donc va bien au-delà des 64 millions que vous demandez madame sénatrice donc même avis. Merci monsieur Savoldelli. merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes, mes chers quand même ce monsieur le rapporteur Jean, j'entends bien, vous nous dites ça va être basculé vers la mission Écologie Monsieur le Ministre, nous parle du fond Vert 300 millions rien à dire là-dessus. Sauf que le fond Vert, c'est pas le sujet qui a été abordé par ma collègue Jourda, qui a fait l'objet de l'unanimité de la commission d'enquête du Sénat du travail du Sénat unanimité donc il faut qu'on aborde cette question il y a des coups de dépollution à faire, moi je vais vous dire il y a un problème de santé publique, je vous apprends rien, on se retrouve les uns et les autres sur tous nos territoires à découvrir des molécules qui sont dangereuses dangereuses dans les sols, vous savez tout ce qu'elles peuvent rejaillir dans l'air ou dans l'eau ou les deux en même temps, et moi je vais vous dire j'ai vécu une situation et je la vis toujours dans mon département, catastrophique, je pourrais les collèges il y en a un qui a empêché l'ouverture à Ivry-sur-Seine, traces de mercure laissées par une fabrique de lampes Philips on a retardé plusieurs années un collège désarmer ouvert à Vitry sur Seine, sans parler du collège Saint-Exupéry à Vincennes, fermé depuis déjà 5 ans après, découverte d'une pollution aux solvants chlorés Tétra Chloro éthylène, le département a d'ailleurs sollicité plusieurs fois le fond de recyclage des friches du plan de relance pour avancer sur la dépollution, donc faut pas confondre voyez le fond qu'on propose pour le monter à un niveau de 75 millions avec l'abondement de 64 millions qu'on voterait là

on est preneur, hein, certes, mais on n'en a pas été là, donc voilà, je voudrais vous dire que là, il faut à mon avis qu'on prenne les les mesures nécessaires, il y a un enjeu pour les communes, les départements et les régions, c'est que on pourra pu aménager. Et alors encore moins acquérir des surfaces pour réaliser des projets pour nos populations. Donc, plutôt que d'occuper des espaces naturels de de dégrader la nature de certains sols, il faut arriver à dépolluer ses sols et leur donner une nouvelle affectation et avec l'utilisation des des matériaux faire esprit de responsabilité merci. Merci monsieur Savoldelli Madame Jourda. Merci madame la présidente, simplement il faut que les choses soient bien claires à un certain moment donné lorsque nous établissons donc des rapports qu'est ce que nous avons constaté, on a constaté que l'amalgame n'apporte rien, qu'on ne peut pas mélanger les fonds, c'est pour ça que nous souhaitons des fonds spécifiques, la dépollution étonne âgé, c'est un enjeu de de santé publique et lorsqu'on aura pas un tiré à part qui permettent on a évalué 75 millions d'euros, mais pourquoi pas, que sur une année, on l'a évalué en l'lycée avec les financements voulu sur 10 à 12 ans parce que la situation est catastrophique et si nous voulons apporter de la calotte de vie et de l'environ et qui soit digne, aujourd'hui, de ce qu'on peut attendre, c'est pas par par le Fonds Vert c'est pas par pas, par ces procédés là mais c'est par le fait de positionner budgétairement chaque fois des des fonds spécifiques dépollution nous y tenons et franchement c'est pas ce que c'est une question de salut public, tout simplement, c'est pas une question de vouloir dépenser et quelque part, on sait bien qu'on ne s'y trouver un moment pour le quoi qu'il en coûte des fonds, il faut les trouver pour la dépollution parce que on a une loi sur l'eau, on a une loi sur l'air et je rappelle que pour les sols nous sommes orphelins d'un outil législatif, ce que nous présidons nous préconisions dans notre rapport d'ailleurs. Merci, cher collègue, s'il n'y a plus de prise de parole, je mets aux voix cet amendement 56 rectifié bis qui a reçu 2 avis défavorables qui est. On compté

Qui s'abstient, il n'est pas adopté Alors, le 205 rectifier et il est présenté par. Madame Cohen. nous souhaitons inclure les salariés dépendant des Centres de santé du régime minier dans la prime Ségur ces derniers qu'il s'agisse des soignants, des intervenants à domicile ou des personnels des laboratoires de biologie en sont exclus, il ressort de cette inégalité de traitement des difficultés de recrutement pour les structures, mais également une perte relative de gain de pouvoir d'achat, à travail égal, le régime minier à travers son offre de soins, encadrés par filière, il est régulièrement contraint dans ses Budgets du fait d'une volonté ancienne d'extinction du régime, si la crise sanitaire a fait la démonstration de son utilité en étant l'acteur prioritaire, voire unique sur des pans entiers du territoire donc du Pas-de-Calais, il n'en demeure pas moins que l'action sanitaire et sociale de l'Agence nationale pour la galerie garantie des droits des mineurs, a dû se contracter, faute de budget adapté, filière il l'Agence nationale pour les garanties des droits des mineurs, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ont évolué et s'adresse aujourd'hui à tous les assurés sociaux, sur les anciens territoires miniers limiter les moyens en ne prenant en compte que la population des assurés du régime minier crée donc une situation de tension sur les ressources, les personnels participe, pour l'essentiel au maintien à domicile des personnes âgées, au travers des soins coordonnés médico-sociaux nous travaillons régulièrement avec les salariés de ce régime et le représentant, développer l'offre de soins est devenue un impératif de santé publique et de lutte contre la désertification médicale, c'est aussi une mesure de justice sociale, en particulier pour les aides à domicile, qui accuse des rémunérations plus faibles que leurs collègues faute d'inclusion dans le Ségur l'objectif donc de cet amendement et de corriger cette inégalité et d'offrir au régime minier, les moyens de son développement, je vous remercie. Merci madame Cohen avis de la commission. C'est manifestement un amendement d'appel comme tout à l'heure, puisque là encore, on ne peut pas s'il y a pas d'autorisation d'engagement, on ne peut pas avoir de crédits de paiement mais j'entends le message en même temps c'est un peu difficile de pouvoir répondre sur un certain nombre de sujets en. Je dirais, en essayant de le greffer sur le plan de relance donc une demande de retrait. Si Monsieur le Ministre. Même avis pour compléter les personnes en question ont déjà bénéficié du Ségur de la santé par par des de complément mensuel et puis évidemment ce genre de mesures devrait être adopté en cas du PLFSS c'est pas dans le cas du PNF donc demande d'Europe. Merci, monsieur le Ministre, je mets aux voix l'amendement 205

nous allons procéder au vote des crédits de la mission, plan de relance figurant à l'étape et je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission je vais donc mettre aux voix, les crédits de la mission et j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe, les républicains sur les crédits de la mission, plan de relance, je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

plus personne ne demande à voter Le scrutin est clos.

les crédits sont adoptés, nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission investir pour la France 2030 figurant à l'état B. 8 amendement faisant l'objet d'une discussion commune le 122.

les auteurs de cet amendement, souhaite que les comités stratégiques de filières puissent être soutenus dans le cadre de la mission investir pour la France de 2030, ces comités stratégiques permettent en effet, concrètement, de faire valoir et de rapprocher les attentes objectifs et intérêts des différentes composantes de grands domaines d'activité, les CSF doivent ainsi devenir des leviers essentiels dans la mise en oeuvre d'une planification dont les objectifs sont définies en concertation avec le Parlement n'étant doté d'aucun budget propre les CSF dépendent des composantes qui dispose des moyens les plus importants, au 1er rang desquels les organisations patronales cette dépendance financière tend à favoriser les projets portés par les plus grosses structures au détriment de projets structurels collectif issu de la coopération entre acteurs ce temps pourtant, ces projets qui mériteraient d'être particulièrement soutenus merci. Merci monsieur seulement le 121 rectifier Il est défendu. 121 rectifié. Merci madame la présidente, cet amendement, un objet ambitieux et indispensables accélérer la reconstruction de l'hôpital public au fil des séances dans cet hémicycle sont évoqués lors des débats budgétaires, lors des questions au gouvernement, l'état de l'hôpital public, les conditions de travail, la réouverture des lits et services l'amortissement de l'inflation, la reconnaissance de la pénibilité et bien d'autres enjeux. Aussi, pour mettre fin plus rapidement à des taux de vétusté gravissime, suite à l'effondrement des taux d'investissement depuis de trop nombreuses années, nous vous proposons donc d'accélérer transférer 200 millions d'euros vers un nouveau programme intitulé plan de reconstruction de l'hôpital public au sein de la mission Investissements d'avenir. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre par cet amendement, nous souhaitons donner les moyens à la France de devenir la première économie de la transition en accompagnant les entreprises dans la durée pour transformer en profondeur leur modèle d'affaires, nous sommes vraiment ici dans la transition, l'objectif est d'accompagner pendant 5 ans 40000 PME dont les gestionnaires bien souvent nous ni la conscience des risques que font peser sur elle les instabilités environnemental et social, ni les moyens d'adapter leur modèle, on est ici dans l'adaptation dans un 1er temps des actions telles que bilan scope 1 2 3, calcul de la dépendance à l'environnement comptabilité triple capitale économie de la fonctionnalité écossais éco- conception seront menées, monsieur le Ministre vous avez essayé de me rassurer tout à l'heure, mais je ne suis pas tout à fait rassuré je veux vraiment que la France s'engage dans cette transition et nous, on ne va pas pouvoir continuer dans la techno-science qui a montré l'épreuve de son inadéquation à soutenir le vivant sur cette planète, merci. Merci le 147 rectifié bis madame latex Quentin. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, l'innovation est au coeur de notre économie et vous l'avez évoqué, hein, mais quand on pense innovation on pense souvent, innovation technologique, il est vrai qu'elle est essentielle, innovation procédé l'innovation produit mais si elle est essentielle, elle n'est pas la seule innovation l'innovation sociale, elle aussi, fait progresser les entreprises peut progresser l'économie, l'ESS et porteuse d'innovation sociale c'est le l'article 15 de la loi dite Hamon qui défini l'innovation sociale qui peut être soi qui peut avoir vocation à répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits Se doit de répondre à des besoins sociaux par une forme d'entreprises innovantes, donc cette innovation sociale est vraiment essentiel, elle porte une finalité sociale, une et une éthique ou une fine, une il nous semble important de de porter davantage cette innovation sociale : le secteur de l'économie sociale et solidaire et les associations porteuses d'innovation sociale échappent la plupart du temps au dispositif d'aide aux innovations alors que, comme pour tout type d'innovation, les besoins d'investissement sont importants, y compris en terme de recrutement de salariés donc pour ces raisons, nous souhaitons soutenir l'innovation sociale, en créant un nouveau programme intitulé Aide à l'Union, à l'innovation sociale au sein de la mission Investissements, je vous remercie. PME engagée dans l'innovation pour la bifurcation écologique certes des aides existent, mais elle se concentre sur l'innovation à haute intensité technologique, ce que nous vous proposons : c'est la création d'un outil de soutien à l'investissement dans l'économie du futur low-tech tout aussi crucial pour notre avenir, il pourra concerner notamment des projets d'investissements dans les secteurs du bâtiment, du textile, des emballages de l'agroalimentaire, des mobilités local mais aussi le secteur de l'ingénierie de l'innovation sociale quant aux et aux modalités précises de la part d'investissement matériel immatériel, le niveau de cofinancement requis, cela pourra être déterminée par décret en concertation avec les opérateurs de l'État, de plus, ces activités sont pour une grande part en lien avec leur territoire participant des circuits courts et non délocalisent. Merci le 155 rectifié bis identique madame Blatter ex-. Merci madame la présidente, défendu. Et il nous passons au 123. Monsieur Salmon. la disparition totale des plastiques jetables est programmée pour 2040, une date bien tardive mais qui impose de restructurer la filière industrielle pour le réemploi des emballages 500 millions ont déjà été mobilisés via le plan de relance, les besoins sont estimés entre 1 et 2 3 milliards d'euros, je ne vous apprends rien en disant que l'actualité croule sous ces problématiques de plastique en ce moment, on parle beaucoup des pots de yaourt en polystyrène qui n'ont pas de filière, on fait mine de dire qu'ils vont être recyclés en fin de compte, tout cela finit dans l'incinération dans les sols et dans les mers, je pense qu'il faut agir très rapidement parce que, là aussi, les populations sont en train de gangréner l'ensemble de la planète, comme on en parlait tout à l'heure pour les sols merci. Merci monsieur seulement et il reste le 193, il n'est pas défendu, donc il tombent, nous passons à l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur spécial. Bien, bien, l'amendement 122 qui nous propose un soutien au comité stratégique avec une notation de 200 millions d'euros, un tel amendement ne trouve pas sa place dans le cadre de la mission, je rappelle que le fil rouge, c'est l'innovation, donc c'est une demande de retrait. L'amendement 121 qui propose un plan de reconstruction de l'hôpital public retrait également la démarche fait sens compte tenu de l'état des hôpitaux, c'est d'ailleurs pourquoi certains des crédits de France 2030 sont fléchés vers le médical, l'action de maturation de technologie recherche développement, valorisation de la recherche du programme 424 qui contribue à la maturation des technologies, des dispositifs médicaux numériques et innovant et l'action un financement de l'écosystème de l'enseignement supérieur et de la recherche de valorisation du programme 425 qui soutient la recherche biomédicale, le développement des connaissances en matière de santé, l'amélioration des pratiques médicales notre avant, à travers les instituts et les projets de recherche IHU RH donc retrait, là encore, l'amendement 125 fond de transformation des entreprises à hauteur de 200 millions d'euros, cet amendement ne trouve pas sa place dans le cadre de la mission en dépit du sujet abordé, je rappelle que le fil rouge de la mission, c'est l'innovation, donc c'est une demande de retrait, l'amendement 147, il s'agit là de d'une d'un amendement qui vise à une aide à l'innovation sociale, avec une dotation de 100 millions d'euros, pose une véritable question, celui du financement de l'innovation sociale, je rappelle que le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, a défini d'innovation sociale, comme une réponse nouvelle à des besoins sociaux nouveaux, ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché, les politiques sociales, ces innovations concernent des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le logement, la santé, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, la discrimination, or, France 2030 n'est pas dénué de toute dimension sociale puisqu'une de ses priorités, mieux vivre, il a ainsi pour objectif de placer la France à nouveau en tête de la production de contenus culturels et créatifs de développer une mobilité sobre souveraine et résiliente d'investir dans une image, y a une alimentation saine, durable et traçable tous ces objectifs répondent à des besoins sociaux, souvent mal satisfait je demande donc le le retrait, l'amendement 124 qui tend à créer un fonds de soutien aux TPE-PME d'innovation bifurcation écologique low-tech a donc c'est un sujet pertinent qui ne nécessitent pas la création d'un nouveau programme pour autant l'ADN de la mission, c'est l'innovation, je le répète, la transition écologique représente un des deux des objectifs de la mission quant aux critères low-tech, c'est-à-dire une technologie durable utile accessible encore ce qui importe c'est l'innovation qui est incarné par un projet qui permet de mieux vivre de mieux produire pour rejoindre les priorités de France 2030 donc je propose le retrait sur cet amendement, amendement 155.

à la stratégie de recyclage et réincorporation des matériaux recyclés, une dentiste une dotation de 370 millions d'euros de fonds publics et consacré aussi, tiens, il y avait au soutien de l'innovation pour l'économie circulaire pour la période 2021 2027, complétant ainsi les montants prévus dans le cadre du plan de relance, j'ai en tête d'ailleurs un démonstrateur de recyclage enzymatique des plastiques à Toulouse qui permet de recycler massivement la plupart des plastiques en boucle fermée, donc c'est un avis de retrait. Merci, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le Ministre même même avis. Hé bien, c'est entendu, je vais donc mettre aux voix, ces amendements commençant par le 122 qui a donc reçu de demande de retrait ou avis défavorable.

il n'est pas adopté le 124 et le 155 identique. Ont reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement même vote. Ils ne sont pas adoptés le cent vingt-trois donc même avis même vote il n'est pas adopté, nous allons procéder. Au vote des crédits de la mission investir pour la France de 2030 figurants à l'étape et je vous rappelle que la commission des finances, est favorable à l'adoption des crédits de cette mission je mets aux voix les crédits de la mission sur lesquels je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe LR sur les crédits de l'oncle de la mission investir pour la France en 2002 2030, je vous rappelle que l'avis de la commission est favorable, il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement, le scrutin est ouvert.

a voté, le scrutin est clos à l'heure. Voici les résultats sur les crédits de la mission votants 343 exprimés 343 pour 316 contre 27 les crédits sont. C'est. Nous continuons avec le 119. Madame mon. cet amendement a pour objet de mettre fin à cette situation incompréhensible et indécente qui consiste pour une entreprise à toucher des aides de l'État pour mieux les reverser aux actionnaires en licenciant au passage ces salariés en effet les entreprises du CAC 40 ont rémunéré leur actionnaires à hauteur de 80 milliards d'euros, enfin je le répète, 80 milliards d'euros au titre de l'exercice 2021 et risque de battre ce record au titre de l'exercice 2022, dans le même temps, elles ont annoncé 62500 suppressions d'emplois, dont 30000 en France, pourtant 100 % de ces entreprises du CAC 40 ont bénéficié de larges aide de l'État, sans aucune contrepartie, nous souhaitons donc conditionner les aides de la mission Investissements d'avenir à l'absence de versement indécent de dividendes ou de licenciement non justifié à la faveur de la crise. a un conditionnement des aides de la mission à l'absence de versement de dividendes et licenciements économiques pour les entreprises qui font du bénéfice, ce dispositif n'est pas opératoire, les porteurs de projets sont généralement au stade de l'amorçage aujourd'hui par ailleurs, le dispositif n'est pas cohérent avec la nature même des projets, la prise de risque existe, or celle-ci peut conduire à terme soit la réussite donc naturellement au versement de dividendes, soit l'échec et malheureusement délire sur Simon économique c'est un avis défavorable.

C'est ça. Qui s'abstient, il n'est pas adopté après l'article 43 un amendement 120. Monsieur Salmon. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, à nouveau, un amendement qui a pour objet de mettre fin à une situation incompréhensible, tout le monde convient qu'il est impératif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et le gouvernement nous incite à couper le WiFi à des pulls pour pouvoir baisser le que on doit reconnaître que pour le chauffage dans cet hémicycle, il fait encore bien chaud, comme dans l'ensemble du Sénat le gouvernement, lui, mise sur des technologies qui, dans l'avenir pourrait peut-être répondre à ces enjeux, nous souhaitons donc par cet amendement conditionner les aides de la mission Investissements d'avenir au respect de véritable engagement écologique, l'innovation, qui est le maître mot, ce soir, l'innovation pour l'innovation, la création de nouveaux besoins ont déjà porté leurs fruits empoisonnés, je pense qu'il faut vraiment avoir un regard critique sur toute l'innovation, elle peut être facteur facteur de progrès pour l'humanité, mais également facteur de destruction merci. Merci, avis de la commission, monsieur le rapporteur spécial. a un autre collègue Salmon demande le conditionnement de l'E3, les crédits des crédits de la mission à l'engagement annuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il se trouve que France 2030 a pour priorité la dès qu'il aborde la décarbonation et elle vise à consacrer 50 % de ses dépenses à la pendant décarbonation de l'économie et 50 % % des acteurs émergents porteurs d'innovation sans dépenses défavorables à l'environnement, aucun projet ne peut être sélectionné s'il comporte un impact négatif pour l'environnement, c'est donc une demande de retrait. Monsieur le Ministre. Ma vie, cet amendement est satisfait. Très bien, je vais donc mettre aux voix l'amendement 120 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui s'abstient, avis défavorables. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Mes chers collègues, je vais le. Et la séance prochaine séance mercredi 30 novembre à 10 pour l'examen de la mission Relations avec les collectivités territoriales du projet de loi de finances pour 2023 la séance est levée.